La séance est ouverte.-- Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Nous n'avons pas reçu d'observation.-- Il y en a-t-il en séance.-- Je n'en vois point. Le procès verbal est donc adopté sous les réserves d'usage. Madame, la Première ministre. Mesdames, et messieurs les ministres, mes chers collègues. L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Notre séance et retransmise en Direct sur Public Sénat et sur notre site. Au nom du bureau. J'appelle chacun d'entre vous a observé au cours de nos échanges. Le respect qu'il s'agisse du respect des uns et des autres ou celui du temps de parole. Je vais donner immédiatement la parole au président Patrick Kanner pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame, la Première ministre.-- Ils avaient 23 ans.-- Ils sont morts pendus. Exécutés en public pour l'un d'entre eux par le régime des mollahs iraniens pour crimes de guerre contre Dieu.-- Ils avaient un nom. C'est. Et Majid Reza Rahnavard en leur mémoire. J'aimerais que le Sénat respecte quelques instants de silence. Nous pouvons craindre qu'il ne soit que les premiers d'une longue liste. En effet, le régime iranien a annoncé via une justice expéditive avoir condamné 9 autres personnes à la peine capitale dans le cadre des manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini. La répression s'abat aveugle, violente, sanglante depuis le début de la contestation, plusieurs milliers de personnes ont été arrêtées plusieurs centaines sont mortes, 400 viennent d'être condamnés à des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Les séides du régime veulent écraser un mouvement populaire où les femmes sont en première ligne ou l'émancipation et le but.-- Femme, vie, liberté, ce slogan est porteur des espoirs d'un peuple. Nous devons être à la hauteur de cet espoir. Le 10 novembre dernier, ma collègue Marie-Arlette Carlotti vous interpeller pour demander que la France exige l'exclusion de l'Iran de la Commission de la condition de la femme à l'ONU, malgré le retard, je suis heureux que votre gouvernement fini par écouter cette juste revendication cette exclusion est actuellement en débat à New York. Certes des sanctions ont été prises par l'Union européenne. Certes les condamnations internationales existent mais sont-elles suffisantes. Devant l'ampleur de la répression. Mes chers collègues. Un baril de pétrole vaut-il plus que le sang d'un manifestant. Aussi ma question est simple, alors que le peuple iranien se bat pour les droits humains. Comment la France peut-elle l'aider. Comment la France peut-elle agir au sein de l'Union européenne pour que la répression cessent et que la jeunesse iranienne éprise de liberté, remporte son combat de Lumières contre l'obscurantisme. Pour vous répandre la parole est. Est à madame la Première ministre madame Borne.-- Monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Président, Patrick Kanner.-- Femme, vie, liberté. Ce slogan est née en Iran. Mais il a très vite dépassé les frontières.-- Ces 3 mots sont des symboles puissants et un appel à la liberté.-- En Iran, le régime. Leurs droits aux femmes, il les cibles pour ce qu'elles sont. L'oppression que subissent les femmes ne date pas de la mort tragique de Mahsa Amini. Elle s'incarne dans les lois du pays. Port du voile obligatoire mariage précoce dès la puberté, interdiction de l'avortement crimes d'honneur en Iran devant les tribunaux. La parole est parole d'une femme vaut la moitié de celle d'un homme. Contre la négation de ses droits humains, un mouvement de protestation aînée qui ne faiblit pas. Qui s'est étendu à toute une partie de la jeunesse et se poursuit depuis maintenant 2 mois. Il se poursuit malgré la répression violente qui a fait plus de 500 morts, dont des dizaines d'enfants. Au moins 15.000 personnes ont été arrêtées. 2 Iraniens ont déjà été condamnés à mort et exécuté à la suite de leur participation aux manifestations. Ils se poursuit malgré l'emprisonnement de journalistes toujours plus nombreux. Le président de la République a eu l'occasion de dire notre admiration notre respect et notre soutien à celles et ceux qui défendent les droits fondamentaux en Iran. Qu'il me soit permis au nom du gouvernement, de leur rendre hommage, de leur dire que nous sommes avec eux.-- Face à la gravité de la situation, la France n'est pas impassible. Nous agissons. Monsieur le Président. Un air de manière forte ferme et résolue. Avec nos partenaires européens. Nous avons envoyé lundi pour la 4ème fois un signal puissant d'unité et de fermeté aux autorités iraniennes. Nous avons encore élargi la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives en y ajoutant 20 membres du régime ainsi que la radio-télévision iranienne IRIB. Nous prenons des sanctions significatives. Gel des avoirs, interdiction de pénétrer sur le territoire de l'Union et interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition des personnes et entités concernées.-- Notre ligne est claire, nous mettrons tout en oeuvre pour que le régime, le régime iranien, sorte de sa logique de répression. Nous avons ainsi adopté il y a 2 jours de nouvelles conclusions du Conseil de l'Union européenne sur l'Iran qui établissent un cadre d'action européen d'une grande fermeté. Enfin, nous soutenons les aspirations démocratiques du peuple iranien la Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Catherine Colonna a remis a remis samedi avec son homologue allemande le Prix franco-allemand des droits de l'homme. Ah Mahsa Amini et aux femmes iraniennes. Ces efforts nous les poursuivrons sans nous laisser intimider. Le régime cible nos ressortissants. Certains sont détenus dans des conditions inacceptables. Nous continuons à exiger leur libération, ce qui se trouve en Iran ou envisagent de s'y rendent s'expose à des risques de détention arbitraire. Je veux donc ici renouveler mon appel à la plus grande vigilance. Monsieur le Président. Je le redis, la France est et restera aux côtés de toutes celles et tous ceux qui combattent pour la liberté pour les droits humains. Je vous remercie. Monsieur le président. Madame le 1er ministre. Nous avons ici au Sénat soutenu l'Arménie. Nous avons ici au Sénat soutenu l'Ukraine. Nous voulons aussi soutenir le peuple iranien dans son combat pour la liberté. J'aimerais qu'un jour ce peuple puisse faire sien. Ce beau poème de 1942 de Paul Éluard Liberté, j'écris ton nom.-- Merci monsieur le président. Je vais donner la parole à notre collègue Éric Gold pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole.-- Merci Merci monsieur le président. Monsieur le Ministre, malgré des efforts notables pour le déploiement de la fibre. Il ne se passe pas une semaine sans que les élus locaux soient sollicités pour des dysfonctionnements. Chantier technique abandonné coupures fréquentes liées au réseau aérien travail bâclé sur les raccordements. Refus d'installer le cuivre dans une construction neuve qui bénéficient pas encore de la fibre abonnement prélever sans que l'habitation soit raccordé déception par rapport au débit. Les motifs de ce mécontentement général sont innombrables. L'Arcep vient d'ailleurs de publier les résultats d'une analyse de terrain qui confirment la situation avec des défauts, notamment sur l'état des câblages. Et ce que certains appellent des raccordements en plat de nouilles. Constat partagé par la Vicat présidée par notre collègue Patrick Chaize. Qui dénonce des opérateurs faisant trop souvent appel aux sous-traitants sans vérifier la qualité ni la pérennité des installations. 15 à 20% des abonnés seraient ainsi touchés par un dysfonctionnement. Monsieur le Ministre. Nous sommes encore loin du 100 pour % comme annoncé du territoire couvert par la fibre en 2022 et les chiffres du déploiement cache d'importantes disparités territoriales entraînant pour certaines ou pour certains plutôt une double peine. En effet, en parallèle de ce déploiement souvent insatisfaisant le réseau cuivre et progressivement abandonné et donc mal entretenues, y compris dans les territoires qui n'ont toujours pas la fibre et qui subissent des délais de dépannage atteignant plusieurs mois. Des territoires qui était déjà fragile et qui se trouve davantage pénalisés par cette situation. Avec des conséquences potentiellement critique je pense par exemple à la télé-assistance qui ne peut fonctionner qu'avec un réseau efficient. Monsieur le Ministre, j'aimerais donc savoir comment l'État entend agir vis-à-vis des opérateurs qui n'ont pas tenu leurs engagements. S'il est prévu de mieux informer les élus commune par commune, et de remettre à niveau le service après vente du réseau cuivre qui continue de jouer un rôle essentiel dans certains territoires. Je vous remercie.-- Pour vous répondre. La parole est au ministre délégué en charge de la transition numérique des télécommunications Jean-Noël Barrot vous avez la parole. Le ministre, monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Gold je partage évidemment votre constat con concernant les défauts de qualité dans le déploiement de la fibre qui place nos concitoyens parfois dans des situations intenables, elles sont le fruit de plusieurs facteurs, d'abord la rapidité du déploiement de la fibre dans notre pays en 10 ans, la France est devenue le pays le plus avancé en matière de fibre avec 77% des locaux raccordables deuxièmement l'existence de réseaux de fibre historiquement mal dimensionné notamment ceux qui ont été déployés, parmi les premiers, il y a 10 ans enfin au recours, vous l'avez cité un nombre trop important de niveaux de sous-traitance même si cette pratique a largement diminué face à l'accroissement des difficultés qui remontent de toutes parts, et en particulier de la part des élus locaux. Le gouvernement et l'Arcep ont saisi la filière télécoms afin qu'elle formule des engagements, ces engagements ont été pris fin septembre et s'articule autour de 3 axes Première éléments le renforcement de la qualité des interventions avec une certification des compétences minimales requises pour les raccordements finaux. Oui. Deuxièmement, la transmission par les opérateurs commerciaux de leurs plannings d'intervention et le partage des comptes rendus d'intervention, de manière à ce que les, les pannes éventuelles puissent être secouru plus rapidement. Enfin le 3ème axe et la reprise des infrastructures. Que ce soit au niveau des points de mutualisation des des réseaux vieillissants ou mal dimensionnés. Plusieurs opérateurs ont déjà notifié leur plan de reprise de 1000 points de mutualisation correspondant à 450.000 locaux ce plan, le gouvernement veille à sa mise en oeuvre le contrôle en et on revient à l'Arcep et des points de suivi régulier. Sont effectuées en présence des associations d'élus pour autant le déploiement de la fibre et le projet d'arrêt de commercialisation du cuivre ne doivent pas se traduire par une baisse de qualité de service ou une exclusion de certains de nos concitoyens, la qualité du réseau cuivre doit être maintenue en attendant sa fermeture technique. L'État ne transigera pas et sur ce point, notre message est clair pas dépose du cuivre tant qu'une solution fibre n'est pas proposé aux usagers. Sachez monsieur le sénateur que je veille personnellement à ce que cette transition s'accompagne par ailleurs des garanties nécessaires de disponibilité de qualité et d'abord d'habiliter de service pour tous nos concitoyens. Merci, monsieur le Ministre, je vais maintenant donner la parole à notre collègue Paul Toussaint Parigi pour le groupe écologiste solidarité et territoires. Monsieur le président, Mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Elle porte sur un écocides annoncé que l'État ne peut ignorer par l'ampleur de la menace qu'il fait peser sur notre région. Je parle du projet du centre d'enfouissement de Donka adios aux abords immédiats du 2ème plus grand fleuve de Corse le Tasigna nous classé zone Natura 2000 et zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Ce projet fou, c'est le stockage et l'enfouissement de 120.000 tonnes de terre amiante faire et de 70.000 tonnes de déchets ménagers par an sur 30 années. Un affouillement des sols abyssal dans une zone géologique instable, les pieds dans l'eau, où d'importants glissements de terrain ont déjà été observés espère géologue hydro-biologiste confirme et signe le risque majeur de destruction de cet écosystème. Aux conséquences dramatiques sur la santé humaine et les générations à venir. Je rappellerai ici que le Tasigna nous irrigue toute la plaine orientale ou une grève qui ont la agriculture diversifiée de qualité labellisée est connu mondialement pour sa production d'agrumes est un inestimable réservoir de biodiversité au coeur même duquel INRA et Cirad abri d'un précieux conservatoire génétique des agrumes d'Europe et d'ailleurs mettre en péril l'alimentation en eau potable de toute une région. Détruire le coeur agricole de la Corse hypothéquer la santé humaine des générations futures. Voilà Monsieur le Ministre, les enjeux dont il est question. Un acte criminel en devenir dans la scène se joue aujourd'hui sous nos yeux. Depuis 6 ans. Nous demandons une interdiction totale de ce projet. Malgré un arrêté de refus initial pris par le préfet, Alain Thirion en 2016 et les prescriptions du préfet François Ravier en 2019 pour minimiser les risques du projet le combat juridique continue. Alors ma question est simple, serez-vous au nom du devoir supérieur de l'État à protéger la vie et son écosystème. Être à nos côtés pour interdire la logique mercantile qui hypothèque notre territoire et sacrifie la terre que demain nous lèverons à nos enfants. Je vous remercie. la cohésion des territoires. Monsieur Christophe Béchu. Vous avez la parole. Monsieur le Ministre.-- Vous remercier pour votre question, vous pointez du doigt et vous braquer les projecteurs sur la situation très complexe depuis 2015 de la Corse en matière de gestion de déchets. Un tiers des déchets qui sont produits sur l'île sont triées orientées vers le continent les 2 tiers, soit 160.000 tonnes doit être traité localement. Or les 2 installations de stockage qui existent ne peuvent permettent d'en accueillir que 100.000 tonnes par an. Face à ça une société oriente Environnement a demandé en 2016 à pouvoir stocker le long du fleuve ta vie nous. Sur un site qui potentiellement présente des risques d'affaissement un site de stockage. Le préfet a donc refusé. Sauf que le tribunal administratif a cassé ce refus, en 2020, le préfet a donc pris une décision qui a consisté à limiter avec la vie d'Ineris un stockage partiel et en novembre 2022, le tribunal administratif a exigé que nous donnions une autorisation complète de stockage.-- Ce sujet est évidemment problématique. Il y a l'autorité de la chose jugée et il y a ce que vous décrivez en termes de risques pointés y compris par les autorités préfectorales. Plus largement, c'est la question de la gestion des déchets en Corse qui se pose. J'aurais dû. Il y a quelques jours accompagné le mini Gérald Darmanin à l'occasion d'un déplacement en Corse pour aller rencontrer les élus, puisque ce sujet fait partie de l'agenda des discussions que nous avons avec les élus insulaires, c'est reporté aux premières semaines de l'année 2023. Je ne ferai pas mes responsabilités, j'irai à la rencontre des élus. Je soutiens évidemment la position du préfet. Je soutiens les inquiétudes qui sont exprimées par les élus locaux. Je soutiens les risques qu'ont été pointés par beaucoup d'acteurs, il faut qu'on arrive à trouver une solution. Compte tenu de la décision du tribunal administratif et des risques que vous pointez, nous allons nous y atteler dans les prochaines semaines.-- Merci la parole est à notre collègue Daniel Chassain pour le groupe les indépendants République et Territoires, vous avez la parole. 4 ou 5, c'est la teneur des courriers que nous continuons à recevoir tous dans les ventes des entreprises en détresse sur nos territoires. Certes il y a eu des évolutions sur le dispositif de soutien de l'État aux entreprises mais cela ne paraît pas suffisant pour un bonhomme Nantel au-dessus de 10 salariés nous. Des fermetures dans le futur, la solution réside dans l'augmentation de notre production d'énergie et diversification de nos sources énergétiques, nous venons d'examiner un projet de loi afin d'Aix d'accélérer le déploiement de GNR des ENR pour la une filière nucléaire d'avenir on devrait se prononcer sur une nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie. le 16 novembre dernier, madame, la Première ministre a évoqué un travail prochain dont l'objectif sera, je cite, de relancer rapidement les investissements dans les barrages sans nécessiter une remise en concurrence, qu'en est-il dans de nombreux territoires, notamment en Corrèze. Nous avons un projet de station de transfert d'énergie par pompage steps avec un pompage en en un heure creuse dans la Dordogne redonna ce projet de stockage malheureusement depuis des décennies, il permettrait de répondre aux pics de consommation turbines à la demande et d'éviter de manquer d'électricité. Et de réduire les coûts. Mais voilà, EDF n'est pas en position d'investir dans ce projet en grande partie à cause de l'ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques imposée par l'Europe, pourtant c'est le ministre de l'énergie doit être plus que jamais une question de souveraineté pour notre pays. Monsieur le Ministre où en sont ceux de ses dossiers. Qu'en est-il des discussions engagées avec Bruxelles à quoi. Pouvons-nous nous attendre concernant les demandes de prorogation des concessions. Merci. Pour vous répondre. La parole est à monsieur Christophe Béchu Ministre de la Transition écologique la cohésion des territoires. Monsieur le président, Mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs. Monsieur le Sénateur Chassaing.-- Vous avez bien posé les termes du débat. L'hydroélectricité la première source d'énergie renouvelable dans ce pays avec 26 gigawatts et nous pouvons nous féliciter des investissements qui ont été réalisés par nos grands anciens dans ce domaine mais vous avez raison aussi il y a à la fois une volonté gouvernementale rappeler exprimée par la Première ministre et une situation qui est complexe compte tenu de ses perspectives d'ouverture à la concurrence et plus encore du précontentieux qui a été engagé par l'Union européenne sur l'absence de mise en concurrence pour le renouvellement des concessions d'hydroélectricité.-- La volonté du gouvernement de faire en sorte de favoriser des énergies renouvelables et de nous appuyer sur celles qui ont fait leurs preuves, comme l'hydroélectricité. Je veux saluer le Sénat qui en votant l'article 16 quinquies de la loi d'accélération sur les énergies renouvelables a notamment validé un processus qui devrait nous permettent de contourner cette difficulté puisque cet article prévoit que les dispositions sur les investissements pour assurer la pérennité d'un ouvrage hydroélectrique puisse être réalisée sans mise en concurrence, c'est le chemin que nous souhaitons suivre. J'ajoute que vous avez cité aussi celui dont nous avons besoin EDF la nomination d'un nouveau président directeur général la discussion de sa feuille de route la caractérisation d'une stratégie qui est à la fois celle du gouvernement et celle de l'entreprise avec la perspective de la nationalisation nous permettent d'avoir un alignement d'astres pouvoir relancer ce sujet. La route est semée d'embûches. Mais l'enjeu de la souveraineté de retrouver la maîtrise de notre énergie commande que nous trouvions des solutions, je sais votre attachement à ce sujet, vous l'avez évoqué avec moi dès le tout début du mois de juillet lors de notre première rencontre. Je peux vous assurer que notre détermination est totale pour dépasser ces obstacles précontentieux et relancé ce dont nous avons besoin une production française d'énergies renouvelables qui nous permettent de tenir le choc est d'offrir à nos entreprises et nos ménages des tarifs qui soient compétitifs.-- La parole est maintenant à notre collègue Patrick Chaize pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président. Mesdames, et messieurs les ministres, mes chers collègues. La crise énergétique, nous amène à revoir nos organisations domestique comme professionnel afin d'adapter nos consommations aux ressources disponibles. Vous nous annoncez cependant depuis quelques jours des phases de délestage de réseau. Ces coupures locales limitées dans le temps impacteront l'ensemble des usagers ménages entreprises Service Public. Les réseaux de communications électroniques qui ont pourtant prouvé leur caractère indispensable durant les phases de confinement seront également touchés. Je souhaite donc attirer l'attention du gouvernement sur le cas spécifique des réseaux de téléphonie mobile qui achemine notamment les appels d'urgence. En effet, en cas de coupure même entonné les numéros d'urgence, y compris le 112 ne seront pas accessibles sur des pans entiers de de nos territoires. Je pense notamment aux secteurs moins dense qui se sont desservies que par un seul pylône tout défaut d'alimentation électrique entraînerait alors une impossibilité d'accéder au service. Les antennes n'étant pas considérées comme des équipements prioritaires. De surcroît les éléments les plus structurants du réseau pour être aussi concernés. La coupure de certaines antennes aura des répercussions sur le réseau national. Les opérateurs pourraient être être par exemple dans l'incapacité d'assurer des missions de sécurité intérieure. C'est pourquoi Monsieur le ministre, ma question est double. Quelles garanties pouvez-vous nous donner sur l'acheminement des numéros d'urgence vers les centres de régulation en tout temps et en tout point du territoire. Envisagez-vous de donner un statut de réseau essentiel aux réseaux de communication, je vous remercie.

Permettez-moi monsieur le sénateur. De saluer d'abord l'immense travail des Salia salariés d'EDF qui mettre notre pays sur la bonne voie, ainsi que l'esprit de responsabilité des Français puisque RTE nous annonce une diminution de presque 10 pour. De la consommation électrique la semaine dernière par rapport aux années précédentes dans notre pays. La continuité des appels d'urgence que vous évoquez repose sur le 112 qui a l'Avantage d'être mutualisées entre tous les opérateurs. Nous oeuvrons depuis cet été à limiter au maximum les conséquences d'éventuels délestages sur les réseaux de télécommunications et donc sur ces appels d'urgence. Il s'agit d'un travail inédit titanesque du fait de la nature et des choix historique d'organisation des réseaux en France. Il suppose de déterminer l'impact croiser des 60.000 points d'alimentation du réseau électrique avec les 110.000 équipements télécoms dont 80.000 antennes et 30.000 équipements structurants qui leur permettent de communiquer entre elles. Je rappelle par ailleurs que même en l'absence de les les stages les re-le réseau Télécom n'est pas infaillible et que chaque antenne dans notre pays tombe en panne pour raisons techniques ou en cas d'intempéries en moyenne une fois par an. À la demande du gouvernement, les opérateurs ont ainsi déjà pris des mesures importantes, ils ont renforcé dès cet Automne l'alimentation de plus de 1000 ne est coeur de réseau, en les équipant de batterie supplémentaire je veille à ce que ces batteries soit testé désormais chaque mois ils ont considérablement réduit par ailleurs les délais de transmission de la carte de couverture du 112 afin que le ministère de l'Intérieur puisse déployer des moyens de secours additionnels en cas de besoin. En complément, je vais vous dire qu'en cas de délestage. Nous demandons aux opérateurs de réquisitionner tous les équipements mobiles disponible ainsi que les équipes d'astreinte afin de renforcer la résilience du 112. Nous verrons également à ce que tous les opérateurs effectuent des simulations pour prioriser les antennes à préserver pour renforcer la résilience du 112 sur la balle du travail réalisé cet Automne par les préfets et né disent vous le voyez, Monsieur le Sénateur, le gouvernement est pleinement mobilisée pour garantir l'accès aux numéros d'urgence des Français en cas de délestage mais aussi pour garantir la résilience du réseau Télécom ces prochaines années.-- Monsieur chaises.-- J'entends votre réponse Monsieur le Ministre, je ne nie pas vos échanges avec les opérateurs. Mais reconnaissez qu'ils sont un peu tardif. D'autant que je ne suis pas persuadé que le délestage soit vraiment la solution. Plutôt que des mesures punitives. Je pense que des actions récompense sur les tarifs par exemple pourrait être plus vertueuse. Les territoires ruraux vont être pénalisés. Attention donc à ce que les zones délestées ne soit pas une fois de plus les zones délaissées. La parole est à notre collègue Nathalie Goulet, pour le groupe de l'Union centriste. Oui, monsieur le président, Mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues. Le Parlement européen à la demande du groupe Renaissance et donc de votre gouvernement a obtenu le vote d'un amendement qui fait état de sa préoccupation au vu des subventions versées aux associations liées aux Frères musulmans qui pourraient être mieux contrôlés. Ça pourrait être une bonne nouvelle mais pourquoi proposez-vous à Strasbourg ce que vous refusez ici en effet avec notre groupe nous dénonçons depuis longtemps ces anomalies et je dois dire que le mot est assez faible et notamment lors d'une question d'actualité sur le même sujet au gouvernement le 25 novembre 2021 sans aucun résultat. Plus récemment, le gouvernement a retoqué plusieurs amendements au PLF pour la 3ème année consécutive visant à contrôler les financements des associations. Nous parlons d'à peu près 2 millions d'euros. Quand allez-vous être plus vigilant sur ces financements. Il ne suffit pas de s'indigner de la campagne du Conseil de l'Europe pour la diversité en Europe faisant figurer une jeune fille voilée. Il aurait fallu faire en sorte que cette campagne ne soit pas lancé cette indignation a été veuille véritablement efficace si on en juge l'affiche de la campagne de l'UNICEF que j'ai la, la journée de l'enfant avec une jeune fille voilée voilà très efficace, c'est très intéressant. Donc se préoccuper s'indigner condamné n'est pas suffisant quand allez-vous assécher les financements des Frères musulmans leur interdire tout financement public et les inscrire sur la liste des organisations terroristes. Je vous remercie. La parole est à madame Colonna. Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.-- La protection de nos institutions, contre les ingérences étrangères est nécessaire à l'intégrité de nos démocraties. Cela requiert en effet de la vigilance. Croyez bien que le gouvernement est mobilisé et actif. Pour que les institutions européennes intègre bien le risque de telles ingérences quelle qu'elle soit, je dis bien quelle qu'elle soit et défendent notre socle commun de valeurs. personnellement et avec Laurence Boone. À mes côtés, j'ai personnellement saisi à ce sujet. La Commission européenne et le haut représentant. Il y a plusieurs mois et je l'ai fait à nouveau auprès de Josep Borrell. Mi-septembre, si ma mémoire est bonne. Nous continuerons donc madame la sénatrice de pousser le sujet notamment pour un suivi plus fin des activités des associations financées par l'Union européenne afin qu'aucune d'entre elles ne promeuvent sous sous influence des agendas. À rebours À rebours de nos objectifs d'intégration d'émancipation citoyenne et d'égale dignité entre les femmes et les hommes. L'inscription que vous proposez des Frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes n'est pas possible madame la sénatrice car cette organisation ne répond à aucun des critères fixés par les règles européennes. Cela ne change rien cependant à notre détermination à préserver le bon fonctionnement de notre démocratie française et européenne. Je vous remercie.

bien qu'il gangrène notre République. Ils espionnent nos boîtes nourrissent des think Tang. Je crois vraiment qu'il faut en finir avec cette naïveté et et très franchement exiger de la Commission européenne. Des respon c'est le minimum que nous puissions demander. La parole est à notre collègue Éric Bocquet pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste avait la parole. membres du gouvernement. Chers collègues, le 10 juillet 2018 lors de l'examen du projet de loi. Liberté de choisir son avenir professionnel ici même notre groupe était intervenu à l'article 1er en n'émettant ces critiques, je cite. D'un compte personnel de formation abondé en heure nous passons donc à un compte abondé en euros. Si le nombre d'heures prises en charge par le compte personnel de formation diminue. Il est à parier que les formations les plus longues et les plus coûteuses devront faire l'objet d'un financement complémentaire reposant essentiellement sur le salarié, Dimanche, à l'Assemblée nationale en a adopté un amendement au projet de loi de finances pour 2023 qui prévoit de contraindre les salariés à prendre en charge de 20 à 30% du coût des formations. Nous avions donc raison d'alerter, il y a 4 ans sur les risques de faire peser sur les salariés. Le prix des formations professionnelles. C'est d'autant plus injuste qu'elle est justifiée uniquement et essentiellement par un souci d'économie budgétaire qui est décidément l'Alpha et l'oméga de vos choix budgétaires. Monsieur le Ministre, ma question est double. La subvention de l'apprentissage a coûté 4 milliards d'euros à l'État ce désengagement organiser des entreprises au financement de l'apprentissage vous amène à réduire le droit à la formation de fête. Première question, allez-vous revenir sur ces subventions indues qui oppose, formation professionnelle et continue, des salariés 2ème question allez-vous enfin accroître le contrôle les organismes de formation qui accumule une rente générée par les coûts exorbitants des formations proposées au détriment des salariés de notre pays.-- Pour vous répondre. La parole est à la ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle Madame Grosjean. Il avait la parole. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. J'ai écouté avec attention ce que vous venez dire à l'intention du gouvernement. Et je crois que c'est tout le contraire. Rendre le système plus juste et plus efficace. Combattre les fraudes. Régulariser les dérives et toujours associer davantage la formation un projet professionnel d'avenir et notre ambition.-- Je le rappelle, le gouvernement a porté ces derniers mois un certain nombre de mesures pour améliorer la qualité de la formation. Cela a conduit à éliminer environ 2 tiers des certifications dans l'intérêt n'était pas avéré pour l'évolution professionnelle de nos concitoyens. Il a également conduit à évincer des plateformes les organismes de formation qui ne satisfaisaient pas les exigences attendues. Par ailleurs, nous avons depuis octobre. Débattu et adopté ensemble une loi portée par votre collègue Martin lévrier visant à lutter contre le démarchage abusif et les fraudes. Il s'agit à présent pour y parvenir, de faire en sorte que chaque bénéficiaire s'engage de manière active dans sa formation avec une participation financière. Mais nous voulons que ce soit juste. C'est pour cela que les demandeurs d'emploi en seront dispensés tout comme les salariés qui ont co-construit un projet professionnel avec leur employeur via un abondement. C'est sur ces bases, efficacité et équilibre que vont s'ouvrir les concertations avec les partenaires sociaux avec les parlementaires avec les acteurs de la formation pour déterminer le niveau de cette participation et son plafonnement. Convaincu que la formation est une clé essentielle dans les parcours professionnels et cette responsabilité de l'individu ne doit pas être un frein à l'accès à la formation, nous y serons attentifs. Je vous remercie. Oui, madame la ministre, votre réponse n'est pas rassurante. En 2018, le directeur de cabinet de votre ancienne collègue Muriel Pénicaud disait aux partenaires sociaux qu'il n'y aurait pas de problème de financement, car les cotisations patronales seraient augmentés en conséquence s'il le fallait, en tout cas vous venez nous expliquer que, avec ce choix, c'est la première fois dans notre histoire sociale que nos concitoyens pour devoir financer eux-mêmes l'accès à un droit acquis. La parole est à notre collègue André Gattolin pour le groupe du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.-- Merci monsieur le président, ma question s'allait s'adresse à à Gérald Darmanin. Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur le Ministre de l'ONG Save Gore Defender qui offrent pour la défense des droits humains à l'échelle internationale vient de publier un rapport mettant en évidence l'existence de 110 postes illégaux de police chinois répartis sur plus de 50 pays post-qui viserait à contrôler réprimer voire à extrader hors de tout cadre légal des citoyens chinois vers leur pays d'origine. L'accusation est grave, elle est très grave, mais le rapport en question est étayée par de très nombreux documents et témoignages sur ces pratiques illégales opérées hors du territoire chinois en France. Ce sont pour l'instant 4 postes illégaux de ce type qui ont été dénombrées à pareil Noisy-le-Grand et Aubervilliers, surveillance des établissements taïwanais ouïgours ou Tibétains pressions exercées sur des citoyens chinois réfugié en France contrôle politique de la diaspora. Bref, la liste des activités illicites dénoncée par l'ONG est longue. Interrogé plusieurs responsables chinois ont reconnu l'existence de ces postes en arguant que ceux-ci se limiterait à des services d'assistance de type consulaire auprès de leurs concitoyens. Mais même sans autorisation de telles Optile activités sont de toute façon illégale au regard du droit international au dollar et si les faits dénoncés par l'ONG sont avérés, ce serait sans conteste une atteinte très grave à notre souveraineté et même une forme toute nouvelle de séparatisme opérer sur notre sol par des agents illégaux d'une puissance étrangère aujourd'hui tous les pays européens concernés par cette enquête, à l'exception de la Grèce et de l'eau et Hongrie ont déjà officiellement diligenter une enquête sur ces pratiques inquiétantes. Alors Monsieur le Ministre, avez-vous ou entendez-vous diligenté une enquête de ce type en France. Je vous remercie. Monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. Je veux dire ici, qu'effectivement, la France ne peut accepter en aucun cas des atteintes à sa souveraineté. Entend lutter extrêmement fortement contre les influences étrangères sur son sol et n'acceptera pas. nous ne pouvons accepter dans le passé dans le futur que les règles internationales notamment qui prévoit l'accueil de ces des ressortissants des pays se fasse au détriment de nos bonnes relations entre États qu'il s'agisse. De la Chine et de tout autre État. La DGSI est en effet à l'écoute de révélations qui ont été pu être mises en place par cette organisation nous gouvernementale, elle a d'ailleurs travaillé en amont bien évidemment de ces révélations. Je lui ai demandé d'accentuer évidemment son enquête de renseignements auprès du gouvernement de la République et du président de la République. Vous comprendrez que ce n'pas ici que je pourrais détailler ses résultats mais si vous le permettez, je vous invite à vous rapprocher de la délégation parlementaire. Au renseignement qui elle est sous le sceau confidentiel défense pour que nous donnions toutes les informations. Si le président du Parlement Gérard Larché ou la prison de la semaine nationale délégation elles-mêmes le président buffet venait à demander ces informations. Ce qui est certain c'est que pour tous les. Pays extrêmement agressif. Dans la contre-influence sur notre sol. Le président de la République. Voilà plus de 4 ans a demandé des moyens renforcés. La DGSI j'aurai l'occasion si vous le souhaitez dans le cas de la délégation enseignement de pouvoir les détailler. Pour vous rassurer que la France n'acceptera jamais ce genre de pratiques qui reste à confirmer. Pour ce qui concerne les quatre postes qui ont été évoqués par cette ONG en France. Merci. La parole est à notre collègue Corinne Imbert pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président, ma question s'adressait à madame, la Première ministre pour évoquer notre souveraineté sanitaire car le sujet à la fois économique et sanitaire des pénuries de médicaments et de dispositifs médicaux. Cela fait des années que ça dure. Mais aujourd'hui, le niveau des manquants a atteint des sommets. C'est du jamais vu. Paracétamol et Amoxicilline continue de faire l'actualité et le ministère impose quant à lui des contingentements. Mais aujourd'hui c'est aussi l'un des acteurs mondiaux des industries de santé. Le dernier fabricant français de poches de perfusion pour les hôpitaux qui est en redressement judiciaire et qui cherche un repreneur. Et si aucun repreneur n'est trouvé d'ici le 5 janvier. Alors l'entreprise risque de fermer définitivement les hôpitaux s'inquiète. Il n'avait pas besoin de cela comment demain pourront toujours s'approvisionner en poche de perfusion. C'est un nouveau symbole. Nous, notre indépendance sanitaire qui est en danger. Comment expliquez-vous cela. Monsieur le ministre et que comptez-vous faire. Pour vous répondre. La parole au ministre de la Santé et de la prévention. Monsieur François Braun.-- Les causes liées à ces pénuries de médicaments sont multiples. Déjà la crise Covid augmentent une modification de prescription, plus 13% par exemple pour le paracétamol.-- Il y a également des soucis sur le principe actif et tout l'intérêt de rapatrier ce principe actif en Europe et en France dans le cadre du plan France 2030 par exemple également des soucis de production ou de ou de distribution comme s'est récemment le cas concernant le Doliprane pédiatrique qui est produit essentiellement en Allemagne et avec un mouvement social chez Sanofi qui heureusement a pris fin récemment et qui va nous permettre de retrouver nos stocks. Cette situation vous le savez n'est pas propre à la France, elle concerne l'ensemble du territoire européen, voire plus. En ce qui concerne l'Amoxicilline c'est une pénurie au niveau national il y a un défaut de production. Notre système de surveillance qui est porté par l'Agence nationale du système du de sécurité pardon du médicament nous permet de choses nous permet déjà d'être alerté très tôt puisque les alertes arrivent lorsque nos stocks diminuent en dessous de un mois pour la plupart des produits donc ça veut pas dire que nous n'en avons plus en tout cas, les stocks sont extrêmement bas et elle nous permet aussi d'identifier les causes ces causes nous permettant d'avoir des actions ciblées en fonction du médicament ces actions ciblées. C'est l'interdiction d'exporter pour les grossistes lorsque les médicaments sont en France c'est une distribution plus équitable sur le territoire national via là aussi des grossistes répartiteurs. C'est une prescription avec en officines pharmaceutiques la possibilité de donner ce dont on a besoin, voire même de des conditionner les boîtes.-- Nous travaillons aussi avec les sociétés scientifiques pour pouvoir. Travailler sur les alternatives puisqu'il n'est pas envisageable. Bien entendu que nous ne puissions pas traiter l'ensemble des Français et puis vous le savez, France 2030 et le programme qui va nous permettre de ramener en France les productions ont tout du moins en Europe pour faire de la France un produit, un un pays souverain. En ce qui concerne nos produits de santé pour cela. L'agence de l'innovation en santé a été dotée d'un budget plus que conséquent comme vous le savez, je vous remercie. Monsieur le Ministre, merci vous votre réponse. Mais vous n'avez répondu que sur les pénuries de médicaments, vous n'avez pas aborder la question des difficultés de ce fabricant français le dernier fabricant français de poches de perfusion. Mais c'est révélateur. La pandémie a déjà révélé que la fusion de l'Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires avec d'autres agences pour former public Santé publique France. Nous vous avez fait perdre à l'époque toute capacité d'anticipation d'une crise sanitaire. Vous avez voulu une filière française de masques, cela risque de virer à la déroute vouloir retrouver notre indépendance sanitaire bien sûr évidemment nous y sommes favorables. C'est nécessaire et indispensable notamment dans le cadre du contexte international, mais commençons par ne pas perdre celle qui nous reste, c'est l'exemple de ce fabricant de poches de perfusion mais c'est aussi l'exemple de l'Établissement français du sang qui aujourd'hui est en difficulté et qui mérite toute l'attention du gouvernement et si Monsieur le Ministre des hôpitaux ont une dette vis-à-vis de l'Établissement français du sang. Je ne veux pas que notre système de santé soit sacrifiés sur l'autel de Bercy mais si je vous vois monsieur. Non, je ne sais pas la tête, c'est la réalité, ça a été confirmé ce matin en audition par la commission des affaires sociales. Les les pénuries sont insupportables et toute perte de notre indépendance sanitaire. Monsieur le président. Et merci pour le temps serait inacceptable. La La parole est à notre collègue Corinne Ferré pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le Président Madame la Ministre pour répondre aux difficultés qu'il a lui-même créé le gouvernement vient par voie d'amendement au projet de loi de finances 2023, d'instaurer un reste à charge pour les salariés qui mobilisent leurs comptes personnels de formation sur le fond, tout d'abord les Français qui utiliseront leur CPF pour financer une action de formation à nos copains Mans vers la VAE ont un bilan de compétence se verront désormais appliquer une franchise seuls de possibilités d'exonération du ticket modérateur sont prévues en somme. On est très très loin de ce que vous nous si on vend sur vendiez en 2018 avec la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel lorsque vous prétendit et je cite, vouloir libérer les salariés et leur offrir plus de droit, il faut le dire, s'en est fini du CPF dispositif construit par les partenaires sociaux en vue de permettre aux salariés d'établir leur parcours professionnel. Votre mesure est totalement injuste et viendra éloigner encore plus de la formation les salariés aux petites rémunérations et qui sont souvent ceux qui ont le moins accès les mêmes que vous voulez faire travailler jusqu'à 65 ans et donc faire payer pour se former et rester dans l'emploi. Quant à la forme on ne décide pas comme ça un week-end en pleine nuit de remettre en question la formation professionnelle, ceci à coups de 49.3 sans avoir échangé avec les partenaires sociaux alors que ces derniers vous ont remis très récemment des propositions concrètes. Madame la Ministre vous engagez-vous enfin à les écouter en vue de mettre en oeuvre des mesures justes de régulation du CPF qui permette de concilier équilibre financier et développement des compétences.-- Pour vous répondre. La parole est à la ministre déléguée en charge de l'enseignement. Et de la formation professionnelle. Alain Grandjean. Merci, merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice. De quoi s'agit-il. Il s'agit de revenir à l'esprit du compte personnel de formation. D'abord en impliquant davantage les bénéficiaires du compte personnel de formation dans leurs choix de formation pour en faire un acte réfléchi lié à un projet professionnel. Cette disposition, elle s'intègre dans une logique globale, je le disais tout à l'heure elle est portée par le gouvernement depuis plusieurs mois et vise à corriger des dérives et des fraudes. Relatives au système de formation professionnelle des dispositions dont le Parlement a déjà eu à connaître et à débattre ont d'ailleurs été adoptée. Pour cela, nous nous sommes également inspiré. Des propositions faites dans votre propre rapport. Concernant la soutenabilité. Financière de France compétences corédigé avec vos collègues. Frédérique Puissat et Martin lévrier visant à mettre en place un reste à un reste à charge au compte personnel de formation. Pour ces raisons, le gouvernement a déposé début novembre en première lecture à l'Assemblée nationale un amendement visant à mettre en place un mécanisme de régulation du compte personnel de formation pour attendre la fin des négociations avec les partenaires sociaux. Vous l'avez modifié au Sénat pour poser directement le principe d'un reste à charge et le gouvernement a souhaité proposer en seconde lecture un amendement d'équilibre qui pose le principe de participation du titulaire mais aussi de cas d'exonération pour les demandeurs d'emploi et en cas d'abondement par l'employeur dans les formations qui sont proposés. C'est donc sur cette base aujourd'hui que les concertations vont s'engager avec les partenaires sociaux, les parlementaires, les acteurs de la formation pour s'assurer que la participation de la personne ne constituera pas une barrière à la mobilisation des droits. Je vous remercie. Madame la sénatrice. Madame le Ministre je ne voudrai pas être désagréable mais je sais très bien ce qu'il y a dans notre rapport sénatorial. Et vous ne pouvez pas dire ce que vous venez de dire est déformée nos écrits. Non, nous n'avons pas évidemment. Et décidément les mêmes valeurs, car pour moi, le dialogue social c'est la concertation, c'est l'écoute c'est l'échange et des recherches de solutions avec les partenaires sociaux. Une fois de plus, vous avez fait les choses sans eux alors qu'ils ne sont pas opposés à des mesures permettant d'améliorer le système actuel, où est la justice sociale dans ce que vous imposez nulle part, vous ne voulez rien qu'on se co-construire vous voulez obliger les salariés à tirer un trait sur leurs droits sociaux et à payer pour se former. La parole est maintenant notre collègue. Isabelle Raimond Pavero pour le groupe Les Républicains, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Depuis la mort de Mahsa Amini aux mains de la police des moeurs parce qu'elle ne portait pas correctement son voile. Le vent de révolte qu'il souffle sur l'Iran ne faiblit pas et malgré la férocité de la répression, le cri, femme, vie, liberté résonne toujours plus fort dans les rues du pays. Ah ces 3 mots qui incarne tout ce que la charia tente d'étouffer depuis 40 ans, le régime des mollahs réagit de la seule façon qu'ils connaissent par la brutalité, la terreur, la reprise des pendaisons publiques vient rappeler au monde la barbarie à laquelle le pouvoir iranien est prêt pour se maintenir en place les témoignages poignants recueillis au Sénat lors d'une conférence organisée en soutien au peuple iranien ont montré à quel point la violence faisait partie de la nature profonde de ce régime, malgré tout, ils sont toujours aussi nombreux, femmes et hommes a continué de braver la peur a levé pour briser les carcans imposés par la révolution islamique à se battre pour des valeurs qui sont aussi les nôtres et dont nous prétendons régulièrement les défenseurs. La France comme l'Europe reste dans une forme de retrait de moins en moins compréhensible à aux condamnations de principe et au message de solidarité envers le peuple iranien n'ont ainsi ce qui ce que d'une surprenante faiblesse madame la Ministre concrètement quelles initiatives le gouvernement entend-il prendre pour apporter un soutien au soulèvement populaire iranien. Et pour accentuer la pression internationale sur les dignitaires du régime iranien. Merci. Pour vous répondre, la parole et que la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, madame Colonna. Il a dit épuisée. Monsieur le président, Mesdames. Et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Raimond Pavero. Oui, le mouvement de protestation en Iran se poursuit. La répression violente se poursuit également avec. 500 morts, dont des dizaines d'enfants. On a vu aussi avec. Horreur. Des premières exécutions et lundi, lundi, les ministres des Affaires sur étrangères des 27 pays de l'Union européenne ont demandé l'arrêt immédiat de ces exécutions. L'exécution de manifestants ne peut tenir lieu de réponse aux aspirations de la jeunesse. C'est une évidence. Madame, la Première ministre l'a rappelé, la France continue d'agir de manière résolue, il n'y a aucun retrait aucun recul, madame la sénatrice. Un nouveau train de sanctions européennes a été adopté lundi. Qui cible notamment. La police des moeurs, impliqués dans la répression des manifestations. Ainsi que la radio-télévision iranienne. Il ne peut y avoir d'impunité pour les responsables des violations des droits fondamentaux et vous savez que c'est la 4ème fois que les Européens cet automne adopte des sanctions contre l'Iran et ils continueront si nécessaire.-- Ils ont aussi adopté lundi. Pardonnez-moi. De nouvelles conclusions du Conseil très complète sur l'Iran, qui constitue un cadre d'action d'une grande fermeté par ailleurs face à la politique qui est actuellement menée par la République islamique d'Iran nous utiliserons pleinement ce cadre à madame le Première ministre vous l'a indiqué. Par ailleurs la France votera en faveur du projet de texte portant exclusion de l'Iran de la commission des droits de l'homme, des droits de la femme dont font Aux Nations-Unies. Je l'avais indiqué. En audition à la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale la semaine dernière et je vous le confirme. La France voteront en faveur de ce texte. J'ajoute que celui-ci devrait être adopté aujourd'hui même nous continuons d'agir en soutenant résolument cette pulsion de vie qui se manifestent en Iran. Je vous remercie.-- Madame la Ministre, l'Iran est face à un tournant de son histoire la France, l'Europe, la communauté internationale doivent se mobiliser. Il est temps qu'elle se montre à la hauteur du courage des manifestants iraniens notre pays. Fidèle à son histoire et à ses valeurs doit être à l'avant-garde. C'est ce que nous ont demandé au Sénat les résistants iraniens. Merci. La parole est au président Laurent Lafon pour le groupe de l'Union centriste. C'est le ministre de l'Intérieur, il y a quelques semaines, vous annonciez ici même au Sénat que des festivals devront être annulés durant l'été 2024 à cause des jeux olympiques. Cette annonce a provoqué de nombreuses réactions d'incompréhension. La semaine dernière avec plus d'une trentaine de sénateurs et sénatrices, membre de la commission culture, éducation et communication du Sénat, nous avons publié dans le journal Le Monde une tribune pour dire que le JO ne peuvent se faire au détriment des nombreuses. Manifestations sportives, culturelles, festives qui ont lieu traditionnellement partout en France. Madame la Ministre, de la Culture a dans une interview publiée. Aujourd'hui dans le journal Le Parisien précisé que des solutions avaient été trouvées pratiquement avec les tous les grands festivals en tout cas ceux qui recourent aux unités de forces mobiles Néanmoins, de nombreuses questions demeurent. Quid des grands événements festifs qui ont lieu dans un certain nombre de régions françaises durant l'été je pense en particulier au Sud-Ouest de la France avec des fêtes comme celle de de Bayonne ou ou de Quid de la surveillance des plages qui jusqu'à présent sont telles que sur et par des CRS quid enfin des nombreux événements qui, pour se tenir ont besoin des de recourir au aux sociétés de sécurité privées, on le sait les JO vont massivement faire appel à ces sociétés, plus de 15.000. Postes doivent être créés pour faire face aux seuls besoins des Jeux olympiques. Ces sociétés pourront-elles couvrir à la fois les besoins des événements en province et ceux liés aux Jeux olympiques et dans ces conditions, monsieur le Ministre, pourquoi ne pas compléter le dispositif en recourant à l'armée.-- Pour vous répondre. La parole est au Ministre de l'Intérieur monsieur Gérald Darmanin.-- Oui, monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Président la font les Jeux olympiques. À Paris, c'est une fois par siècle.-- Et les Jeux olympiques à Paris avec une cérémonie d'ouverture en dehors d'un stade, c'est une fois tous les 3000 parce que personne ne l'a jamais organisée en dehors d'un stade. Et je pense qu'on peut constater ensemble l'intérêt général qui a de réussir. Je vous en particulièrement sensible, je le sais. Les Jeux olympiques de Paris et les Jeux paralympiques, qui s'étalent durant l'été 2024. Je serai prêt d'ailleurs qu'en 2024 c'est aussi le 80ème anniversaire du débarquement de Normandie, c'est qui. Au mois de juin également il y aura énormément. des forces de sécurité intérieure pour protéger l'ensemble de ces grands événements avec tous ces chefs d'État et bien sûr cette grande miniature à Paris ce que nous avons proposé avec la ministre de la culture avec la ministre des Sports, chargée Jeux olympiques ce n'est pas l'annulation des événements c'est leur décalage notamment dans le temps et je crois que nous avons été en partie entendu. Par exemple, le Tour de France qui ne va pas arriver en 2024 à Paris. Et le 28 juillet mais à Nice le 21 juillet. Voilà quelque chose qui nous paraît conforme à l'intérêt général et conforme à la volonté d'avoir évidemment un Tour de France 24 ou le festival des Vieilles Charrues. Je peux aussi parler du festival d'Avignon et d'autres grands festivals dont Madame, la ministre de la culture à l'occasion d'évoquer un décalage de date pour les Vieilles Charrues. Elles se dérouleront du 11 au 14 juillet au lieu du 18 au 21 juillet. Comme quoi il les on ne capable dans notre pays de discuter en concertation avec tous les acteurs du monde sportif et culturel du monde festif en général pour que ces événements se tiennent mais dans des conditions où on doit comprendre qu'il faut 45.000 policiers et gendarmes pour les Jeux olympiques de Paris de sa de nature jusqu'à sa fin. En ce qui concerne l'armée elle est déjà très largement mobilisés. Si nous l'armée ne tenait pas, par exemple, le site qui ferait partir les bateaux sur la barre, je serai 30 UFM que nous serons obligés d'utiliser par les forces de l'ordre, l'armée, c'est aussi ce qui garde la politique aérienne sous l'autorité de la Première ministre et les luttes anti-drone ou contre l'arrivée de d'avion par exemple au dessus de nos événements. Mais l'armée n'est pas fait pour le maintien de l'ordre. Voilà plus d'un siècle, que nous avons de spécialisée, cela grâce à un certain nombre de policiers. Et de gendarmes. Ce n'est pas pour les confier à la va-vite faut qu'aucun des militaires. On aura l'occasion d'en parler. La sécurité privée. En fait le ministre de, du travail un certain nombre de démarches très positif qui lui permet d'être confiant dans la présence sécurité privée partout sur le territoire national. Merci Monsieur le Ministre pour ces éléments de réponse. Je. N'avons pas forcément compris la façon dont la la la question des festivals avait été abordée jusqu'à présent, vous faites une annonce et quelques semaines après, on nous annonce que finalement les solutions ont été trouvées, dont acte. Et tant mieux, mais pour éviter que ces solutions ne se reproduise. Nous souhaiterions notamment que au niveau des territoires et avec les élus locaux, nous fassions vous fassiez un inventaire précis des manifestations et que vous abordiez concrètement quelles solutions peuvent être trouvées trouvées dans un contexte on le sait et vous l'avez rappelé, qui est exceptionnel avec les difficultés que peuvent engendrer l'organisation d'une manifestation aussi importante que celle des JO néanmoins le dialogue avec les élus locaux sur ce point, nous sommes extrêmement important. Merci la parole est à notre collègue Béatrice Gosselin pour le groupe Les Républicains. Monsieur le ministre, monsieur le président, mes chers collègues mieux chez moi mieux pour ma planète, voici le slogan qui présente MaPrimeRénov aider au financement des travaux de rénovation énergétique calculé en fonction des revenus et du gain écologique des travaux. Travaux principalement d'isolation et de chauffage qui doivent être effectués par des entreprises labellisées Hergé. Lorsque votre logement est mal isolés ou équipé d'un mode de chauffage, dont le coût augmente de façon exponentielle. Vous êtes évidemment intéressés par ce dispositif. Quand vous cliquez sur le site vous lisez une aide accessible à tous propriétaires ou copropriétaires occupants ou bailleurs qui s'adapte à la situation de chacun et favorise des rénovations ambitieuses. Cela paraît simple et attractif. dans dans de nombreux cas pardon les démarches aboutissent et les primes sont versées dans un délai raisonnable. Certains dossiers connaissent des difficultés importantes et les aides arrivent tardivement jusqu'à 10 mois après les travaux. Numéro national 08 injoignable difficultés pour accéder à l'interface dossier accepté dans un premier temps puis refusé pour l'usager c'est 15 jours maximum pour compléter ou corriger un dossier mais des semaines sans réponse de la part du service MaPrimeRénov. Ainsi de nombreuses personnes se trouvent en difficulté financière quand les travaux sont à payer et que l'aide notifiée par l'état se fait attendre. C'est aussi le cas de d'entreprises et d'artisans RGE qui remplissent les dossiers pour leurs clients et qui attendent longtemps les paiements des primes fragilisant ainsi leur trésorerie même des référents en préfecture ont des difficultés à avoir des retours des dossiers en souffrance. Alors Monsieur le Ministre que comptez-vous faire pour améliorer ce dispositif et ne pas mettre, particuliers et entreprises en difficulté.--

Vous avez raison, il existe un certain nombre de dysfonctionnements, mais je crois d'abord qu'ils ne doivent pas masquer l'et 1,5 millions de chantiers qui ont été réalisées dans le cadre de de ma prime rénovent. 1,5 millions de chantiers qui ont qui ont été en particulier et des 80% de ménages modestes et quand on interroge les ménages. 66% des ménages qui ont fait ces travaux n'aurait pas fait ses travaux sans sans MaPrimeRénov néanmoins oui des difficultés existent d'irrégularités d'irrégularités, voire de fraudes ont été constatées et ça nous a obligé dans la volonté du gouvernement d'être très attentif à ces fraudes, de prendre un peu plus de temps sur l'évaluation des de c'est tous les services de l'sont extrêmement mobilisés pour régler ses différends difficultés prendre des contacts individuels avec les familles dans lesquelles les dossiers prennent trop de temps, j'étais avant-hier je crois un rendez vous avec la défenseure des droits et nous avons évoqué un certain nombre de cas qui lui avait été remonté nous travaillons d'arrache-pied pour régler ses problèmes. C'est tout le sens de ce grand service public qui est France rénovent que nous allons faire progresser, que nous allons faire améliorer en termes de performance parce que oui un certain nombre de nombreux travaux ont déjà été réalisés, mais il faut aller plus loin dans la performance et dans des travaux globaux aller plus loin dans les travaux dans les copropriétés dans l'habitat collectif, parce que c'est, oui vous avez raison, comme c'est indiqué sur le site le chantier du siècle et je peux vous assurer de la détermination de mon ministère du gouvernement et de la Première ministre sur ce dossier. Merci. J'entends bien Monsieur le Ministre, mais il est vrai que certaines entreprises rencontrent des difficultés de trésorerie, quand elles ont 15, 20.000 euros pour des petites entreprises c'est beaucoup et je pense que l'Anaes qui est le locuteurs pourrait entrer dans le dispositif du bouquet de France service qui permettrait à à des habitants de pouvoir avoir une réponse rapide et efficace. Merci. on ne fait pas de commentaire sur le commentaire ici. Alors j'ai de la parole maintenant à. Notre collègue Jean-Jacques Lozach. Pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci monsieur le le président, ma question s'adresse au ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires et porte sur la mise en oeuvre de zéro artificialisation nette à l'horizon 2050 et sur la réduction de moitié d'ici à 2030, du rythme de consommation des espaces naturels agricoles et forestiers. Si nous ne contestons pas les objectifs de sobriété foncière et de préservation environnementale de cette réforme structurante pour nos territoires des points de crispations demeurent portant à la fois sur la méthode employée largement descendante et sur le fond des dispositifs. Cette première étape Dusan s'est opérée dans la plus grande confusion générant incompréhension et inquiétude chez beaucoup d'élus. Le Sénat s'est à nouveau saisi de cette problématique en lançant une mission conjointe de contrôle. La proposition de loi issu de ces travaux doit permettre une évolution rapide du cadre juridique Dusan et dans son déploiement de tendre vers davantage de discernement de pragmatisme et de bon sens. Nous attendons ainsi du gouvernement des engagements clairs sur la temporalité avec la révision du calendrier des modifications des documents de planifications sur la gouvernance une grande partie des élus demeurent écarté des négociations, ce qui est inadmissible. Je rappelle que de nombreux départements restent totalement ou partiellement dépourvu de Scott schéma de cohérence territoriale. D'où l'absence d'élus siégeant à la conférence régionale des sera Il faut renforcer la concertation entre régions Scott et bloc communal en dotant le d'une gouvernance plurielle partagée et décentralisée sur la différenciation en garantissant la prise en compte des particularités du monde rural et les spécificités territoriales et fort projet développement local spécificité des zones littorales et de montagne pour préserver le droit à construire des communes rurales, ne faut-il pas laissé à la libre appréciation de leurs élus une surface minimale garantie par le Scott. Enfin la logique Dusan étant celle d'une densification de l'habitat. Que pensez-vous de l'opportunité de lancer un programme national et complémentaire de réhabilitation du bâti ancien en centre-bourg.

Je pense qu'entre la première question au gouvernement à laquelle j'ai eu l'honneur de répondre dans cet hémicycle sur Lausanne au mois de juillet et aujourd'hui je dois être rendu à presque une trentaine d'heures d'échanges avec la chambre haute sur le sujet et la dernière en date à l'invitation de la présidente Valérie Létard. Juste avant que la présentation de la PPL et lieu aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs groupes nous avons même échangé ensemble il y a peu de temps sur le sujet. J'ai rencontré les associations d'élus, et j'attends dans les 1000 qui viennent la fumée blanche du texte que le Sénat va proposer pour faire en sorte d'amender le dispositif dans l'esprit d'ouverture, que le gouvernement a indiqué depuis le début du mois d'août quand il a suspendu la mise en oeuvre des décrets de la fin du mois d'avril. Je vous rappelle les étapes qui sont calés pour ce qui relève du pouvoir réglementaire la réécriture des décrets est prévue pour le début de l'année prochaine. Nous avons fait travailler les agents d'urbanisme et les associations de maires pour déterminer la granularité la manière d'aller écrire ce qui relève des espaces naturels et agricoles. La Première ministre a eu des mots extrêmement clair en clôture du Salon des maires à la fois sur les grands projets d'envergure nationale et sur la garantie rural, ce qui nous importe. C'est d'abord de rappeler et je ne doute pas, compte tenu de vos propos que tous nous sommes convaincus de la nécessité de la sobriété foncière.-- Nous ne pouvons pas continuer à un rythme d'artificialisation qui bouge Nonda phréatiques qui créent des îlots de chaleur et qui nous empêchent demain de préserver des espaces agricoles dont nous avons besoin, y compris pour notre souveraineté alimentaire dans le même temps.-- Il nous faut mieux associer les élus. Parce que dans la façon dont le texte a été rédigé dans les mises en Oeuvres qui sont envisagées, il suscite aujourd'hui des inquiétudes. Certaines sont fondées. D'autres ne le sont pas. Le meilleur exemple c'est que des milliers de communes sont déjà en situation de zéro artificialisation nette sans le savoir, ou qu'elle soit en zone inondable ou qu'elle soit cerné par des AOC ou qu'elle soit au RN eu donc je me réjouis du fait qu'on aura très vite l'occasion de débats non plus du principe mais des modalités.-- La parole est à notre collègue Marc Laménie pour le groupe Les Républicains. Merci. Monsieur le président, madame, la Première ministre Mesdames et messieurs les Ministres ce chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre délégué chargé des Transports et concernant le volet ferroviaire et l'ensemble aussi des personnels. Le 14 novembre dernier, vers 19h, dans les Ardennes à Donchery commune d'un peu plus de 2000 habitants située sur la ligne SNCF, Charleville-Mézières, Sedan, un père de famille et sa fille ont été tuées happée par un train de marchandises en descendant d'un TER qui dessert cette gare ce drame qui a suscité beaucoup d'émotion. Dans ce bourg centre et dans les Ardennes met en évidence les problèmes de sécurité. Cette gare située sur l'axe Calais-Bâle le double voie électrifiée n'est pas équipé de passage souterrain de monde formulée de longue date. Par le maire et ses collègues ni de passage supérieur, seuls des pictogrammes indiquent la présence. D'un train croiseur pour les voyageurs. À noter que cette gare est utilisé aussi par des travailleurs qui font partie d'une section des autres. Sur l'ensemble du réseau national plus de 900 traversée de voix. Pour piétons existe. Monsieur le ministre. Quelles mesures envisagez-vous pour la sécurité du sujet j'ai et, surtout, en parlant de moyens humains, renforcer les moyens humains de présence dans les gares. TER notamment et présence indispensable des contrôleurs. Parce que là malheureusement il n'y avait pas de contrôleurs, ainsi que dans les gares. Je vous remercie. Pour vous répondre. La parole est comme ministre déléguée. Chargée des transports. Seul ministre.-- Monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Laménie. Je veux d'abord m'associer à la motion que vous avez relayée dans l'hémicycle après le drame de Don Cherry. Il y a quelques jours qui a emporté la mort de de de personnes et je tiens à vous indiquer que même si nous n'avons pas encore l'ensemble des éléments sur les causes et conditions de ce drame. Le Bureau enquêtes analyses dans sa section chargée des transports terrestres a ouvert à ma demande une enquête et tous les éléments seront évidemment communiquer le plus rapidement possible après l'ensemble des investigations nécessaires. Cela pose la question d'un certain nombre d'aménagements d'information de formation qui doivent être. Au sein de la SNCF notamment dans des petites gares ou des Alpes, comme c'était le cas en l'espèce j'ai demandé en effet au président de la SNCF au PDG de SNCF voyageurs de prévoir un ensemble d'actions renforcée au-delà de ce qui a déjà été engagé depuis maintenant 3 ans sur la signalisation sur l'information en gare sur la formation des conducteurs sur les points de danger particulier en terme de visibilité ou les difficultés de visibilité. Je suis prêt à regarder le dossier de Don Cherry spécifiquement avec vous mais malheureusement ces quelques centaines de lieux qui sont concernés, encore en France aujourd'hui, nous avons fait un travail engagé par Élisabeth Borne lorsqu'il était ministre chargé des Transports pour aménager un certain nombre de passages à niveau. Mais la question a notamment dans les haltes ferroviaires d'un certain nombre d'aménagements de formation et d'information doivent être renforcées. Je suis prêt il travaillait avec le Sénat, avec vous en particulier, je connais votre engagement au-delà de ce drame sur la question ferroviaire je me tiens donc à votre disposition.

moyens humains, parce que les moyens humains sont réellement indispensable s'il y avait eu un contrôleur je pense que ce drame aurait été évité. J'ai aussi en mémoire. Bah de drames qui ont été évités grâce aussi au personnel et aux conducteurs. Ben un train qui déraille à cause d'un convoi exceptionnel et puis un TER qui avait heurté aussi quelques années un convoi exceptionnel donc merci sincèrement et puis c'est surtout c'est un combat collectif, merci. Merci. La parole est à l'autre collègue Olivier nous pour les groupes de l'Union centriste. Merci monsieur le président, madame, la Première ministre, mesdames, messieurs les Ministres, chers collègues, ma question concerne les ZFE zones à faibles émissions une idée européenne séduisante mais dont l'application est particulièrement complexe et j'y vois une incohérence environnementale une injustice sociale une fracture territoriale voire générationnel et un choix industriel incertain une incohérence environnementale faire peser sur le seul citoyen automobiliste la responsabilité du réchauffement climatique ou ou des particules dans les villes m'apparaît excessif il faudra pas longtemps avant qu'on dise que le responsable du réchauffement climatique. C'est la mobylette de l'ouvrier. La justice sociale. Eh bien ce sont les plus modestes qui sont impactées. Il suffit d'aller dans les quartiers pour constater que vous voyez des véhicules dans les quartiers de de gens modestes et véhicules de vignette cinq des vignettes IV une fracture territoriale voire générationnel. ce sont les habitants des campagnes, ceux de la ruralité du péri-urbain. Ainsi, un couple de retraités qui a une Clio. Diésel depuis plusieurs années ne peut plus aller voir ses enfants en ville et enfin un choix industriel incertain. L'industrie automobile européenne n'est pas prête à cette mutation vers. Véhicules électriques aussi rapidement hein il y a 30% de de de de cette industrie qui est qui est

Monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. Et permettez-moi de revenir d'un mot rapide sur l'objectif des zones à faibles émissions parce qu'elles ne sont pas en soi une volonté évidemment d'exclure de priver d'accès à nos centres urbains toute une partie de la population. Elles viennent d'une nécessité constaté et votée par le Parlement dans deux textes législatifs. Il y a quelques années. La loi d'orientation des mobilités. La loi climat résilience qui vise à mettre en place progressivement, j'insiste sur ce point dans 43 métropoles françaises de plus de 150.000 habitants des zones en laissant une très grande flexibilité aux collectivités locales concernées. C'est un outil entre les mains des collectivités locales concernées qui doit être adapté à la réalité de chacune de ces métropoles et ces agglomérations le calendrier n'est pas très défini, sauf pour les métropoles qui sont en dépassement de normes de qualité de l'air, nous faisons ça précisément pour réduire les impacts sur les qualités sur à l'améliorer et pour éviter les plus de 45.000 morts chaque année, constater à cette pollution. C'est cela l'objectif. En laissant ce trek dans l'flexibilité cette flexibilité s'étend aussi au type de modalités de circulation d'accès qui sont des qui sont décidés pardon par chacune de ces collectivités avec une grande différenciation qui sera précisée est définie par chacune des métropoles le rôle de l'État, c'est d'être en accompagnement pour que précisément les risques que vous identifier à juste titre socio-générationnels ne se réalise pas. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déployé progressivement en lien avec les métropoles des aides pour que la mise en place progressive des ZFE se fasse le mieux possible les elle s'est notamment l'acquisition de véhicules le bonus écologique. La prime à la conversion. Nous avons décidé dans le projet de loi de finances pour 2023 soumis au Sénat et à l'Assemblée d'augmenter à 7000 euros le bonus pour les ménages les plus modestes. Nous avons aussi et c'était une idée de plusieurs sénatrices et sénateurs d'expérimenter une, un, un prêt à taux zéro dans de zones à faibles émissions et de métropole. Aujourd'hui nous sommes prêts à l'étendre et en regarder les modalités avec vous dans les prochains mois. Donc, nous devrons évidemment renforcé encore nos accompagnement travailler avec les métropoles mais je le dis la flexibilité du dispositif est entre les mains des collectivités pour que ça se passe le mieux possible dans le calendrier le plus adapté possible. Monsieur Hulot. Oui, merci Monsieur le Ministre, je ne doute pas évidemment de votre bonne foi de votre bonne volonté, mais ceci dit 3 observations il faudra pas longtemps avant que les ZFE deviennent des zones à à forte exclusion. Je pense aussi que il y a dans cette écologie culpabilisante. Il y a une obsession de la com. Plutôt qu'un souci du bien public et puis aussi un mépris social c'est quand même la France des clopes et du diésel qu'on regarde encore de haut et il y a dans tout ça, un germe de gilets jaunes, je vous remercie. remercie. Mes chers collègues. Madame, la Première ministre. Mesdames, et messieurs les ministres, mes chers collègues. J'ai le plaisir de saluer la présence de la tribune d'honneur. Une délégation de 6 parlementaires de la Chambre des conseillers du royaume du Maroc, présidée par le Docteur Mohamed. Guido, président du groupe d'amitié. Président Président du groupe d'amitié Maroc-France à la Chambre des conseillers, notre collègue Christian Cambon, président du groupe d'amitié et présent à leurs côtés. Lors de l'entretien que nous avons eu. En fin de matinée, nous avons évoqué les principales étapes de leur séjour ici à Paris et en Normandie. Qui leur permettront de s'entretenir avec le ministre Olivier. À la veille d'ailleurs d'un déplacement au Maroc, madame la Ministre, de Madame la Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Il devrait ensuite découvrir les travaux de recherche. Développement menée par EDF en matière nucléaire et d'énergies renouvelables et visiter les chantiers navals à Cherbourg. Cet accueil témoigne de la relation privilégiée qui nous lie. Au royaume du Maroc et à sa chambre des conseillers et de notre attachement à une amitié ancienne qui, dans sa dimension parlementaire s'exprime avec une force particulière, même lorsque quelques tensions a pu apparaître dans la relation bilatérale. Nous avons su garder. Cette capacité d'écoute et de dialogue qui est la marque des amitiés sincères. Le jumelage en cours entre nous assemblées. Et aussi le Sénat italien et le dynamisme des relations entre le groupe d'amitié respectifs. Semble. Une parfaite illustration. Madame, la Première ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues permettez-moi de souhaiter à nos amis, membres de la Chambre des conseillers du Maroc la plus cordiale bienvenue au sénat de la République française. Nous en avons terminé mes chers collègues. Avec les questions au gouvernement. Nous nous retrouverons pour les questions au gouvernement en début d'année avec bonheur. Ce qui me permet de souhaiter à chacune et à chacun d'excellentes fêtes de fin d'année à remercier les collègues, les milices mais ça n'est pas terminée 16h. 35. Nous reprenons pour l'examen d'une commission mixte paritaire. La séance est donc suspendu.

La séance est reprise. En application du 5ème alinéa de l'article 13 de la Constitution ainsi que de la loi organique numéro 2010 tirer 837 et de la loi ordinaire tirer 838 du 23 juillet 2010. Prise sous. Pour son application. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a émis lors de sa réunion de ce jour un avis défavorable, 10 voix pour, 16, ou à contre à la nomination de Monsieur Boris Ravignon à la présidence du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur.

Merci madame la présidente. Monsieur le ministre et ce président de la commission des lois, mon cher collègue, rapporteur. Loïc Hervé, mes chers collègues. Ne boudons pas notre plaisir. Le projet de loi dont nous discutons de manière ultime, que vous avez longuement préparée. Monsieur le ministre. Et mûri après le Beauvau de la sécurité qui a été fortement enrichi par. Notre débat lors de son 1er passage au Sénat est une bonne loi. Qui a réuni une très large majorité dans les 2 chambres du parlement autour de la forte augmentation des moyens engagés pour nos forces de sécurité intérieure. L'Assemblée nationale lors de son examen du texte a retenu une grande partie de nos apports et les a prolongé. C'est donc logiquement que nous sommes parvenus à un accord lors de la commission mixte paritaire. Je voudrais saluer l'esprit qui a prévalu lors de nos échanges avec mon collègue Loïc Hervé bien sûr mais avec notre homologue de l'Assemblée nationale. Florent Boudié, cet état d'esprit a permis d'aboutir à une solution qui préserve. Pour l'essentiel les dispositions que nous avions adopté au Sénat. La commission mixte paritaire ainsi entériné les la plupart des modifications proposées au rapport annexé par les deux chambres. Il me revient de vous présenter les grandes lignes du texte qui présentation qui sera complété par mon collègue Loïc Hervé, avec ce texte. Le ministère de l'Intérieur bénéficiera de 15,3 milliards d'euros supplémentaires pour les 5 années à venir, ce qui lui permettra de nos forces de sécurité, les moyens d'assurer leur mission, moyens supplémentaires dans la première traduction se trouve dans le projet de loi de finances pour 2023, sur les 3 objectifs principaux du texte qu'ont longuement été explicitée par le ministre au Sénat ne nous étions attachés à garantir pour nos concitoyens. L'accessibilité des démarches et le bon accueil. Par les forces de sécurité, nous avions également prêté une attention particulière modalités de répartition et d'installation des 200 nouvelles brigades de gendarmerie et aux concertation indispensable que vous avez démarré. Monsieur le ministre avec les élus locaux. J'y étais donc j'en témoigne l'ensemble de ces points ont été repris par l'Assemblée nationale qui a également prolongé nos apports notamment pour renforcer la lutte contre la cybercriminalité. Et nous avons donc en commission mixte paritaire décidé de reprendre largement le texte tel qu'il a été adopté par les députés, sous réserve de quelques modifications. L'une de ces modifications essentielles concernés, vous le savez, mes chers collègues, les garanties données pour préserver le rôle de la police judiciaire dans le cadre de la réforme de l'organisation de la police nationale. J'ai donc présenté un amendement essentielle qui reprend ses garanties que nous voulions voir écrites dans le rapport d'orientation comme nous, nous en avions convenu avec le ministre d'ailleurs en première lecture, nous avons choisi de réécrire ces garanties dans un amendement qui a été approuvé par la commission mixte paritaire pour l'essentiel, chaque mot ayant été pesé au trébuchet. Pour obtenir l'adhésion de tout ça. Si nous avons inscrit dans le rapport annexé que dans le cas de cette réforme, les magistrats conserveront le libre choix du service enquêteur que ce service devra rester sous l'autorité des procureurs et des juges lors des enquêtes. Nous avons également à ce prix que les affaires sensibles devrait continuer d'être traités par la PJ enfin avec le développement exponentiel de la délinquance organisée qui dépasse les frontières départementales. Il nous a semblé utile de prévoir des structures zonal sans changer l'actuel cartographie territoriale. S'agissant maintenant des articles du projet de loi visant à adapter les prérogatives dont disposent les forces de sécurité intérieure dans la lutte contre les cybermenaces. L'Assemblée nationale a prolongé nos apports. Et en particulier insisté sur le bon traitement des infractions commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé des données. Nous avions ici un débat important sur l'encadrement des cyber assurance dans l'article 6 qui conditionne le remboursement des pertes et dommages. Nous ne sommes accordés sur un délai de 72 heures qui suivent la connaissance par la victime de l'atteinte dont elle a fait l'objet la CMP a prévu un délai de 3 mois pour l'entrée en vigueur de cette nouvelle obligation, le temps pour les assurés, d'en prendre connaissance.-- Mais nous avons voulu modifier aussi certains des articles additionnels qui avaient été intégrés par l'Assemblée nationale. Nous avons finalement conserver les droits nouveaux d'assistance des victimes par un avocat mais nous sommes en revanche revenu sur les articles 6 bis, 6 bis B et six Bissey qui reprenaient des dispositions l'avait dit si superfétatoire. Nous avons également conserver la demande du rapport sur la protection des collectivités territoriales. Nous nous sommes et des entreprises et leur ville Narbr éviter aux intrusions numérique. Nous sommes en contrepartie tombés d'accord pour supprimer la plupart des autres rapports confirmant conformément à la jurisprudence traditionnelle du Sénat.-- Concernant l'amendement que j'avais présenté relatif à l'amélioration de la réponse pénale sur les violences faites aux élus les refus d'obtempérer, les rodéos urbains, à l'Assemblée nationale. À tout à fait suivi notre point de vue là même. Enrichi avec des peines complémentaires permettant de rendre plus efficace. Ces sanctions, je m'en réjouis. La réduction commune du texte que nous vous proposons d'adopter aujourd'hui me semble équilibrée, efficace à la hauteur des enjeux auxquels doit faire face, police, gendarmerie et sécurité intérieure et nous attendons donc avec sérénité. Un vote positif à la hauteur des nouveaux enjeux de sécurité auxquelles nous devons désormais faire face. Je vous remercie. Merci monsieur le rapporteur. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente, monsieur le président de la commission des messieurs les rapporteurs mesdames et messieurs les les sénateurs. Ainsi se termine le long chemin de la loi de programmation et de modernisation du ministère de l'Intérieur. Je voudrais remercier très profondément. L'ensemble des sénateurs qui ont contribué à l'élaboration de ce texte. Je pense comme vous l'avez souligné, monsieur le rapporteur, que c'était un texte co-construit avec le Parlement, avec les deux chambres du Parlement. Je voudrais d'abord saluer le votre, votre travail et ainsi que celui de de Loïc Hervé, je crois d'ailleurs que le lien que vous avez pu avoir avec les rapporteurs de l'Assemblée nationale. Je pense particulièrement à à Florent Boudié évidemment. On était un lien constructif. Me semble-t-il et que le gouvernement n'a rien à retirer de du texte de la commission mixte paritaire puisqu'il a présenté d'ailleurs aucun amendement. à l'Assemblée, ni au Sénat me réjouir d'abord que nous nous sommes mis d'accord sur le rapport annexé qui prévoit le fonctionnement du ministre de l'Intérieur sur 5 ans dans ses à cette acceptation les plus large nous verrons qu'une partie des crédits que vous allez débloquer ainsi serviront pour le débat. On a, on a eu un écho hier mais également qui permet, je le crois d'avoir la définition de ce que nous voulons faire pendant 5 ans au ministère de l'Intérieur après avoir défini des menaces et y mettre ainsi des moyens budgétaires et humains et expliquer comment on y arrive. je pense que c'est un point important puisque seuls nos amis militaires avaient ce jour de programmation et que le ministère de l'Intérieur. Avaient du mal parfois à répondre au temps long puisque c'est un ministère de l'urgence et que ce temps de l'urgence s'empêcher de donner les moyens aux policiers, aux gendarmes ou pompiers aux agents de sécurité civile aux agents de préfecture de pouvoir répondre non seulement aux problématiques d'aujourd'hui mot pragmatique de demain. Je ne reviendrai pas sur la réforme de la police nationale, notamment de la police judiciaire. C'est bien dans cet esprit. Monsieur le rapporteur, que je vais construire désormais le travail j'ai d'ailleurs proposé, monsieur le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale que je vienne en commission des lois la semaine nationale ou je suis évidemment au total disposition pour qu'une fois que le rapport qui sera rendu par les deux sénateurs Madame Bénureau et Monsieur hein. De même, en parallèle avec le rapport rendu par monsieur Bernalicis et Madame Guévenoux et le rapport rendu par l'inspection générale de l'administration et de la justice avant de prendre les textes réglementaires, puisque vous savez que c'est une réforme entièrement réglementaire, je viens de les présenter à la commission des lois du Sénat pour pouvoir vous expliciter. Qu'est-ce que j'ai repris de ces rapports évidemment échangé avec les rapporteurs avec les sénateurs et pour construire cette réforme de la police nationale, non pas contre des personnes mais pour le service public de la sécurité conformément d'ailleurs je crois au très bon compromis que vous avez su. Définir avec vos collègues de l'Assemblée nationale, le 2ème, sujet sur lequel je voudrais insister, monsieur le président de la commission des lois si j'ai proposé à l'Assemblée nationale. Un comité de suivi parlementaire du texte. Que vous allez sans doute adopter dans quelques instants, c'est-à-dire dès le mois de janvier, je propose que la première réunion se tient d'ailleurs fin janvier vous puissiez désigné dans la pluralité évidemment des opinions. Ici exprimer avec vos amis de l'Assemblée nationale. Une réunion qui pourrait servir tous les trois mois ou à Beauvau où évidemment au Sénat ou à l'Assemblée Julien avec l'ensemble des directeurs d'administration de mon ministère pour vous présenter les tableaux suivi des transformations comment on a acceptent. Ces transformations. Comment les crédits que vous nous. Et qui Et qui sont confirmées dans le PLF serve directement à ce sur quoi je me suis engagé et comment les amendements, notamment de nature parlementaire sont respectées et donc je vous proposerai donc tous les 3 mois de tenir ce comité de suivi parlementaire pour bien suivre la loi de programmation c'est à la fois normal puisqu'on le doit évidemment au Parlement. C'est aussi évidemment pour nous toujours un, un gage de conseil de remarques et peut-être même de correction puisque maintenant que nous allons voter la Lopmi la vie va reprendre ses droits et nous avons tous tendance à à revenir si j'ose dire à notre. Travail quotidien terminer madame la présidente, après cet esprit de de Concorde sur ce texte important pour remercier les policiers et les enjeux, les gendarmes, les agents de préfecture, les sapeurs-pompiers, les formations militaires pour le travail qu'ils font tous les jours de leur dire qu'avec les moyens quasi unanime quasi unanime et même pour ceux qui n'ont pas voté voté la présidente ça si je sais que il y a dans ce texte, un peu de votre coeur. Donc je sais que c'est quasi unanimement, ou en tout cas dans l'esprit, si ce n'est dans les votes que nous soutenons les agents du ministère de de l'intérieur et c'est bien avec cet esprit le rapporteur de Brest a eu la gentillesse de dire que j'ai commencé les réunions de concertation sur les brigades de gendarmerie mais de, d'une manière générale que je le rappelle, puisque je crois que sur la sécurité avec un S de nos concitoyens. chacun a pu dans ce débat parlementaire être respecté. Faire entendre sa voix et accordé au ministre de l'Intérieur. Des moyens très importants qu'il sera j'en suis sûr bien utiliser si vous me permettez cette expression, quel que soit le ministres qui termine le quinquennat du président de la République, je vous remercie. Je rappelle qu'en application de l'article 42 Aline. 12 du règlement, le Sénat statut par un seul vote sur l'ensemble du texte. Nous passons aux explications de vote, des groupes à raison d'un orateur par groupe et monsieur Loïc Hervé, vous avez la parole. Madame Madame la présidente. Monsieur le Ministre, monsieur le président de la commission des lois chers marseillais de presse rapporteur sur ce texte, chers collègues. Comme marché de Bresse. Nous l'a indiqué il y a quelques instants, la commission mixte paritaire du 1er décembre dernier parvenu assez rapidement à un accord sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur en tant que co-rapporteur je me suis plus particulièrement intéressé. À l'article 5 qui est relatif aux réseaux radio du futur puis aux articles 7 à 16 de ce projet de loi. L'Assemblée nationale a amélioré enrichi le texte sans remettre en cause les apports du Sénat, ce qui a facilité nos discussions et l'élaboration d'un texte de compromis concernant le délit d'outrage sexiste. L'Assemblée nationale a souhaité rebaptiser outrage sexiste et sexuelles ce qui correspond mieux à la réalité de cette infraction. Elle a en outre élargi le Champ de ce délit pour qui l'englobe tous les outrage commis à l'encontre d'un mineur, alors que nous avions visé visait seulement les mineurs de 15 ans et plus. La commission mixte paritaire a approuvé cette évolution concernant les assistants d'enquête de l'Assemblée nationale a élargi le vivier de recrutement sans abaisser le niveau d'exigence. Ce qui nous a semblé également aller dans le bon sens. L'assemblée a approuvé l'extension des autorisations générales de réquisition qui allégeront la tâche des procureurs en prévoyant qu'un rapport d'évaluation sera réalisée dans un délai de 2 ans. C'est sur la question des amendes forfaitaires délictuelles que le dialogue a été finalement le plus nourris avec nos collègues députés vous voir sous en souvenez le Sénat avait rejeté la proposition du gouvernement d'autoriser le recours à l'AFD. Pour tous les délits punis d'un nom de prison ce qui correspondait à un total de 3400 infractions différentes en effet si elle convient pour la répression de certaines infractions l'amende forfaitaire ne nous avait pas paru adapté à un si grand non rodées de délit. Soit en raison de considérations. Neil soit parce que une amende forfaitaire ne constitue pas à nos yeux une réponse pénale suffisamment forte. Nous avions donc opté pour une approche au cas par cas, en élargissant, en commission, puis en séance publique la liste des infractions pour lesquelles l'AFD est autorisé. L'Assemblée nationale n'a pas remis en cause notre approche mais l'a voulu aller un peu plus loin ce qui nous a posé un problème pour certaines infractions par exemple le tapage nocturne le refus de se soumettre à un contrôle routier ou encore l'entrée dans une enceinte sportive pour troubler le bon déroulement d'une compétition. Nous avons donc obtenu que la liste soit quelque peu concernant le délit de port d'arme blanche, l'amende forfaitaire n'amende forfaitaire délictuelle ne pourra être appliquée que si l'auteur de l'infraction remet volontairement son arme à l'agent verbalisateur. Nous avons également limiter le recours à l'AFD en cas de récidive. Dans certains cas un passage devant le tribunal ou pas paraît en effet nécessaire. Au total, une fois la loi entrée en vigueur la procédure de l'amende forfaitaire sera applicable à 27 nouvelles infractions et pour six d'entre elles l'amende pour être appliquée, y compris en cas de récidive. J'aimerais à présent évoquer d'un mot, l'article 14 bis qui avait été insérés, par le Sénat, l'initiative 2 autres collègues Pierre-Antoine Levi avant d'être supprimée en commission à l'Assemblée nationale. Un compromis a été trouvé qui maintient l'esprit de la mesure, mais en la recentrant sur les seules menaces de mort. Cette disposition qui s'inspire, mon cher collègue des. Remontées des procureurs de la République facilitera les poursuites et nous sommes évidemment d'abord à la commission des lois preneurs des retours des parquets sur ce point. Je termine en me félicitant que la commission mixte paritaire et confirmé notre choix de prévoir à l'article 15, une unité de commandement en cas de crise, en plaçant l'Agence Régionale de Santé, sous l'autorité du préfet et je pense que le Parlement, députés et sénateurs peuvent se féliciter de cette unité de commandement désormais dans la gestion de crise, ça aurait été une des grandes leçons de la crise Covid. Et je pense que les prochaines crises nous montrerons que cela était totalement pertinent. Monsieur le Ministre, je peux ne peut que me féliciter du travail que nous avons eue avec vous-même avec vos services avec nos collègues de l'Assemblée nationale pour arriver à un accord. Cette Lopmi est attendu par nos forces de sécurité. Elles bénéficieront de moyens renforcés, ainsi que de nouveaux outils juridiques pour agir plus efficacement avec Marc il est Daubresse. Nous nous réjouissons, encore une fois, de cet accord important avec les députés et le. Le vote qui a eu lieu à l'Assemblée nationale la semaine dernière parce par son son ampleur montre que cet accord a été encore plus largement soutenu par nos collègues députés que les sénateurs de mon groupe, le groupe de l'Union centriste voteront les conclusions de la commission mixte paritaire et j'invite aussi sur les autres bancs la plupart de nos collègues à en faire autant. Merci. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Jérôme Bureau. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mais sur les rapporteurs mesdames et messieurs les collègues. Permettez-moi de débuter mon propos en saluant le travail des deux corapporteurs ils ont défendu les positions du Sénat en commission mixte paritaire avec conviction et fermeté ce qui a pesé dans notre appréciation du texte soumis au vote aujourd'hui. la disponibilité et la qualité des échanges avec le ministre, je n'insisterai cependant pas trop sur ce point, de peur qu'ils n'utilisent ces compliments dans ces controverses futur avec certains de mes camarades au Palais Bourbon. Je rappellerai d'abord la position initiale de notre groupe. Concernant cette loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur en première lecture nous avions évidemment salué l'effort budgétaire conséquent qui est fait par l'État. Il permettra de répondre aux demandes des citoyens et des élus locaux sur le terrain. relayant quand cela est nécessaire. Ces demandes. Il nous semble cohérent de soutenir la programmation de 15 milliards d'euros. Nous nous sommes félicités des quelques avancées apportées dans le rapport annexé notamment ceux adoptés grâce aux amendements nos collègues. Harribey Jourda et Jacques sur la sécurité civile ou la gendarmerie. Nous avons noté avec intérêt que les recommandations de notre collègue Conconne ont été suivis les dispositions nécessaires à l'application et à l'adaptation outre-mer du PJ. ont été inscrites directement dans la loi conduisant à la suppression d'habilitation du gouvernement à procéder par ordonnances et nous avons évidemment soutenu la meilleure protection des élus face aux violences qui doivent parfois subir j'en profite pour saluer ici le maire de Mont-Cenis en Saône-et-Loire et le personnel de sa commune qui ont eu le malheur de vivre un épisode de menaces de mort la semaine dernière. Tout ne nous allez pas pour autant, même si nous avions voté la Lopmi en première lecture. Ainsi on était-il des AFD dans le Champ a été trop étendu à notre goût. Le texte manque également d'avancer encore sur le rapprochement entre police et population. Je profite de cette tribune pour regretter la suppression à l'Assemblée nationale de l'indicateur de performance budgétaire que le Sénat avait ajouté au PLF à propos des discriminations, commises ou subies par les forces de l'ordre. J'espère que Monsieur le Ministre tiendra sa parole et nous aidera à le rétablir prochainement les discussions sur la police judiciaire ne nous rassurer pas franchement pas plus que les membres d'association nationale de police judiciaire pour parler de manière Hefei mystique je dirais que l'Assemblée nationale ne s'est pas contenté d'améliorer notre texte les discussions CMP était donc très attendue. Elles se sont révélées décevantes sur plusieurs points, le recours aux amendes forfaitaires délictuelles, nous sommes trop développé encore la possibilité de les utiliser en cas de récidive comporte des risques genre retiens cependant que l'AFD été supprimés pour certaines infractions peu compatible avec la reconnaissance des faits qui est au coeur de l'efficacité de cette transaction pénale, je pense notamment au refus de contrôle nous regrettons également les suppressions des articles 6 bis, possibilité pour les victimes de déposer plainte depuis leur domicile ou dans les locaux d'une association d'aide aux victimes, 6 bis B expérimentation expérimentations tendant à la mise en place de brigades de gendarmes et de policiers mobiles ayant pour objectif de recueillir les plaintes des victimes de violences conjugales en territoire rural et 6 bisser droits des victimes à être prises en charge par une personne formée aux discriminations liées à l'identité de genre ou l'orientation sexuelle du positif et malgré tout sorti de la CMP, la suppression de l'article sur la circonstance aggravante en cas de violence gratuite nous semble par exemple bienvenue. Elle donnera moins de travail au Conseil constitutionnel. Je pense enfin aux avancées du rapport annexé qui ont été conservées. Notre groupe se félicite par exemple de la rédaction de compromis trouvé sur la police judiciaire avoir porté les revendications de tous ceux qui ont exprimé leur inquiétude sur la réforme de la police nationale s'est révélé positif, le rapport annexé ne règle pourtant pas tout nous saisissons cependant la balle au bond. Puisque le ministre a proposé après que nous l'ayons demandé à l'Assemblée nationale, la création d'un comité de suivi de notre programmation du ministère de l'Intérieur, vous l'avez réitéré tout à l'heure Monsieur le Ministre, nous lui demandons d'inscrire le suivi des moyens budgétaires de la police judiciaire. Au programme de ce comité de suivi pour conclure le texte sorti de la CMP nous semblent meilleures que sortent celui sorti de l'Assemblée. Il n'est pas fondamentalement différent de celui sorti du Sénat que nous avions voté perfectibles mais attendues par les forces de l'ordre et par nos concitoyens, notamment en ce qui concerne les moyens budgétaires cette Lopmi sera donc votée avec les voix du groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur rapporteur et chers collègues. Le groupe Les Républicains se réjouit du caractère positif de la CMP qui s'est réuni le 1er décembre. Cela faisait en effet plusieurs années que le Sénat a appelé de ses voeux une loi de programmation sur la sécurité. La dernière en date remonte à la loi Loppsi 2 qui prévoyait les moyens pour la période 2011 2013, c'est la fête tout de même 10 ans. Si l'on ne comprend pas bien ce qui a pu contrarier l'adoption de cette le dès le premier quinquennat du président Macron. Nous nous félicitons néanmoins de son adoption imminente Mischa collègue. L'ambition est forte mais la tâche sera rude. Personne ne l'ignore, la France se prépare à accueillir d'importants événements sportifs dont les enjeux en terme de sécurité sont considérables. Qu'il s'agisse de la Coupe du monde de rugby en 2023 ou des Jeux olympiques à l'été 2024, les 15 milliards d'euros supplémentaires budgétés sur 5 ans ne seront donc pas de trop. Nous tenons cependant exprimé de craintes d'une part, il ne faudrait pas que ces moyens viennent à s'évaporer en cours de route, le Sénat sera particulièrement attentif au suivi du déploiement de ses crédits au fil des années à venir et d'autre part il ne ils ne devront pas non plus être happés par les enjeux sécuritaires de 2023 et 2024, les Français auront toujours et encore besoin d'être protégés au lendemain des Jeux olympiques. Par ailleurs, comme a pu le dire le président buffet lors de l'examen des crédits de la mission sécurité du budget 2023, le doublement des effectifs sur la voie publique n'a de sens que si les services traitant les infractions augmentent proportionnellement, et nous y veillerons également. Je ne reviendrai pas dans le détail sur les dispositions du texte. Nos deux rapporteurs, l'ayant fait, dans leurs interventions, je souhaite simplement conclure en formant. Le voeu, Monsieur le Ministre, que la réforme de l'organisation de la police nationale et singulièrement celle de la police judiciaire qui vous occupera particulièrement en début d'année prochaine soit conduite dans le plus grand consensus possible. Pour finir. Le groupe Les Républicains tient à saluer la qualité du travail mené par nos deux rapporteurs Marc-Philippe Daubresse et Loïc Hervé et il est évident qu'une grande partie de notre groupe se prononcera en faveur de ce texte telle qu'issue des travaux de la CMP, je vous remercie de votre attention. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Dany Wattebled. Monsieur

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président. La commission des lois. Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues.-- Je me félicite que la commission mixte paritaire a été conclusive sur un texte concerne l'ensemble l'missions intérieur pour une période de 5 ans.-- ce consensus qui honore nos deux assemblées parlementaires traduit la ferme volonté de la repentance nationale, donner un cadre permettant de renforcer les moyens humains, financiers, technologiques, des forces de l'ordre dans leur mission de protection. relatif à aux questions à la programmation du mystère de l'intérieur. L'attraction ainsi en chiffres et en actes de la considération de la République pour nos forces de l'ordre. Par ce texte nous consacrons une hausse du budget du mystère de l'intérieur de 15 milliards d'euros sur 5 ans. Cette hausse inédite est indispensable pour assurer à chaque instant la sécurité de nos concitoyens face à une délinquance protéiforme fraude trafic. Urbain. Atteintes aux biens et aux personnes. Cette hausse est aussi primordial pour aller améliorer train quotidien des agents du ministère de l'Intérieur et de les rendre plus efficace. Au service et à la production de Français et Françaises. En leur donnant la possibilité de déléguer certains travaux chronophage. tarte, la tâche des forces de l'ordre est immense. Chacun de nous le sait. La délinquance ne cesse de se renforcer. Elle devient de plus en plus violente et également de plus en plus technologique. Oui il y a beaucoup à faire mais ce texte ambitieux. Con si une vérité tellement une première réponse à la hauteur des enjeux. Cette série d'aujourd'hui et de demain. Je me fais ce qui renforce considérablement les moyens humains en créant 8500 postes. Et 200 nouvelles brigades de gendarmerie. Cela permettra de doubler la présence policière sur le terrain. Également, ce texte permet de doter nos forces de sécurité d'instruments modernes grâce au développement d'outils informatiques et numériques. Car moderniser c'est mieux armés. La France et la police. Pour affronter ces nouvelles menaces.

Je pense notamment au cyber attaques contre ce genre de santé qui ne cessent de se multiplier, Villefranche-sur-Saône en 2021. Vitry Le François Corbeil-Essonnes et dernièrement Versailles il y a une semaine. Également satisfait que ce renforcement de moyens de nos forces de l'ordre s'accompagne d'une amélioration de la réponse pénale. Trop souvent, nous avons le sentiment que la réponse judiciaire ne permet pas d'agir sur la délinquance du quotidien. La réponse pénale se doit d'être ferme et efficace.-- Avant de conclure je tiens le salut à cette tribune le courage et le sens du devoir de ces femmes, de ces hommes, gendarmes ou policiers. Qui ont choisi de consacrer leur vie professionnelle et personnelle à la protection de nos concitoyens de nos concitoyens. Monsieur le Ministre, chers collègues. Ce texte propose des avancées qui permettront de répondre aux attentes des forces de l'ordre. Jamais connu depuis. De nombreuses années. Pour répondre à la lutte contre la criminalité, une cruauté qui bien sûr c'est développe sur le nouveau terrain. Ce texte prend également en compte légitimes exigences de nos concitoyens qui aspirent à une plus grande sécurité. Vous l'aurez compris, le groupe les indépendants voteront en faveur de ce texte. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Guy Bénard

Bonjour, madame la présidente. Monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, chers collègues. Nous voici réunis de nouveau pour aborder la trajectoire que doit prendre le ministère de l'Intérieur et les moyens que nous souhaitons lui a loué ce texte avait pour particularité de nous présenter au travers du rapport un accès à son article 1er une vision portée par le gouvernement de la sécurité de la tranquillité publique pour les prochaines années. Nos prises de parole et nos propositions ont permis à notre groupe de défenseurs. Projet pour la sécurité de notre pays a projet cohérent. Ce qui marque le plus dans ce texte, c'est la continuité d'une politique qui se veut plus répressive que protectrice cet aspect. Ne doit pas à ce point négligé la porte. Hausse du lien avec les citoyens la nécessaire confiance de tous envers les forces de l'ordre. l'ordre. À également l'autre aspect essentiel de la prise en compte de l'immense souffrance au travail de nos forces de l'ordre. Nous avons pu exposer le partage. L'objectif du de police bénéficiant de meilleures conditions d'une meilleure formation avec des moyens financiers, humains mobiliers immobilier satisfaisant dans le but d'exercer ses missions auprès de la population auprès de la population mais avec la population et pour la population. Oui, nous soutenons l'action de la police républicaine dans ce qu'elle est au service de toute la population aussi bien les Français à l'aise avec le numérique comme les 13 millions qui souffrent d'électronique L'accès égal pour tous aux services publics, y compris de la police doit prévaloir et l'accueil ou l'interaction avec un agent formé doit rester une option pérenne. Alors d'accord avec vous Monsieur le Ministre, pour de meilleurs équipements pour les forces de l'ordre qui est clairement exercent leurs fonctions dans des conditions matérielles souvent insuffisantes, voire indécente. Comme le rappelle mon collègue Thomas Dossus. Nous alertons cependant sur l'idée d'un policier augmenté. Policiers du équipée oui mais augmenté à quel coût et pour quel but. Nous regrettons que ce texte n'ait pu permettre également de discuter du besoin d'une modification de la doctrine du Mathias de l'ordre en particulier de l'usage du LBD de drone de lacrymo de la tactique de la Nasse ou d'autres techniques d'interpellation que nous jugeons dangereuse. Nous, regrettant qu'aucune réelle et sérieuse avancée sur la réforme de l'IGPN n'ait pu sortir de ce texte, le besoin de sécurité des citoyens portent aussi sur la transparence de l'action de la police, une meilleure gestion des dérives parfois violentes. Une nouvelle vision de l'IGPN mais aussi sur la transparence des données de la police de leur publication de leur transmission est en train de leur transmission aux élus locaux.-- Cette réforme de l'IGPN nous paraît bien plus nécessaire et plus attendues par nos concitoyens que celle dite de la police judiciaire. Se rappeler que le citoyen est au coeur de tout, telle a été notre boussole costaude nous regrettant que malgré le soutien exprimé par le gouvernement sur ces bancs, aucune avancée aux propositions pour généraliser des mécanismes ayant fait leurs preuves par exemple les agents de liaison LGBT plus ou par exemple pour exploiter au mieux les formations nécessaires d'agents formés au cyber harcèlement n'ait été retenue par le Sénat ni par la commission mixte paritaire. Nous regrettons que la prise en compte des droits de la défense que nous portions alimenté par le rapport de la Cncdh de syndicats de la magistrature ou des avocats n'est hélas pas toujours trouvé une oreille attentive comme par exemple dans l'inscription de l'interdiction de la reconnaissance faciale. Mais nos inquiétudes sur les droits des justiciables n'ont pas été dissipé par nos discussions relatives à l'amende forfaitaire. Un outil utile, certes de manière comptable voire cyniquement mathématiques mais dont l'efficacité sur la réponse pénale n'est que peu étudier l'opportunité de poursuivre, qui revient d'habitude au juge et nié de nouveau son application à des infractions autour des stades par exemple semble être une réponse qui n'est pas calibrée face aux difficultés de gestion subie lors des événements du Stade de France par exemple. Et n'y voyez pas un reproche à nos forces de l'ordre. Son utilisation semble très très très variable selon les territoires. Cette mise à l'écart du monde judiciaire. Seule réelle réflexion sur le continuum police justice nous paraît être une erreur. Penser la police sans la justice est une erreur. Bon la sécurité sans les acteurs au coeur des territoires est aussi une erreur. Nous sommes d'accord avec vous sur le poids de la nécessité d'argumenter, les moyens des forces de l'ordre. Nous sommes cependant désaccord profond sur la façon de les employer au mieux. Nous avons soutenu l'augmentation du budget à l'article D E. Nous aurions aimé pouvoir être plus entendu dans nos propositions d'amélioration des conditions de travail des forces de l'ordre de l'amélioration de leurs relations avec les usagers. Notre groupe a cherché à apporter plus d'avancées dans les conditions de travail, par exemple sur leur accompagnement, par des psychologues ou la sanctuarisation des formations au tirs et vous êtes sécurité des citoyens portent aussi sur leur origine en en. C'est pour ça nous avons de nouveau proposé sans succès d'pour le développement d'une réelle police environnementale comme si il y a des par Jacques Fernique les gardes champêtre s'exerçant au sein de la brigade verte par exemple, devraient être clairement distingués des autres services. vous insécurité sécurité des citoyens au niveau local porte aussi sur la gestion des risques incendie amplifiée par l'inaction climatique du gouvernement et nous remercions les parlementaires d'avoir conservé la proposition de notre collègue Monique de Marco sur les besoins du 2ème basses pour les Canadair, nous aurions aimé pouvoir discuter d'autres mesures ou de vision tout aussi importante sur la gestion des frontières par exemple mais en conclusion, j'ai pu à mettre aux prises avec mes collègues rappeler combien les forces de l'ordre sont au coeur de notre pacte républicain, ce sont elles qui endosse le rôle de protection de notre population et doivent assurer la tranquillité publique les crêpes que nous avions exprimées or malheureusement été confirmé les modifications apportées par la majorité sénatoriale n'en fait que les applis fiez l'orientation du ministère de l'Intérieur présenté validé par cette CMP ne nous paraît ni convaincant ni justifiée. Nous ne pouvons donc pas nous y associer. Et nous attendons. Voteront ce projet de loi.

Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ce projet de loi arrive à sa conclusion après. Un parcours législatif et un travail législatif sérieux et méthodique. Je crois que c'est une satisfaction de pouvoir le constater. Cet aboutissement positif doit beaucoup outre naturellement à nos vastes mérite mais à toute la concertation ample et transversale qui l'avait précédé et qui a été menée, je crois de façon sincère et de bonne foi et qui nous a permis de mieux nous informer sur les choix ajouter.-- Le projet adopté met donc en oeuvre. Des. Intentions de des des objectifs d'intérêt public majeur que je veux souligner l'amélioration de l'accueil du public. le renforcement de la lutte contre la cybercriminalité qui savons tout ça péril. Croissant. La lutte plus efficace contre les violences intrafamiliales et sexistes. Et la proximité, l'effort sur le territoire, aussi bien commissariat que brigade. Je crois que ce souci a été bien exprimé par le ministre et nous le nous le partageons. Dans les volumes de de crédit qui sont prévues dans cette programmation, il y a des outils techniques d'avenir aussi bien pour l'émission d'enquête que pour les interventions en particulier à travers le système. Radio futur. Qui sont donc. Nous semble-t-il les bons objectifs. De manière transversale. Les apports de cette loi et j'en ai cité quelques-uns doivent apporter doivent signifier de réels progrès dans les conditions de travail. Des personnels et dans leur sécurité. Ce que nous savons bien que l'émission auxquelles ils font face quotidiennement avec notre soutien moral sont à la fois éprouvante et dangereuse et nous tenons absolument à ce que la poursuite de la vie professionnelle des agents se fasse avec une motivation avec un sentiment d'être soutenus. Par leur hiérarchie et par. Et par les autorités publiques parlement et gouvernement. Et il me semble que ces, ces éléments de progrès qui sont implicites mais qui sont contenues dans le dans le projet de loi, ce sont des éléments très importants. Nous saluons aussi bien sur les mesures d'efficacité introduite dans la chaîne pénale et qui ont été bien délibérée entre les membres du gouvernement déjà et on sait que c'est pas toujours. et entre les 2 chambres du Parlement avec une participation très larges donc il nous semble que les améliorations qui seront apportées à toute une série d'actes de procédure. Vont profiter en effet à l'efficacité de. La mission de, de rétablissement de de la paix publique. Et. Je veux souligner mon tour le le bon choix d'équilibre qui a été fait après mûre délibération quant à la liste des cas où s'appliquent les amendes forfaitaires pour des délits ou pour lesquelles effectivement c'est une sanction adaptée et et qui ne pose pas de problème d'équité ni de de droits de la défense et nous savons bien que dans le dispositif à la fin il y a toujours la possibilité pour la personne sanctionnée de revenir à un traitement judiciaire si elle le préfet.-- Donc nous allons contribuer, bien entendu. Vous savez, pas de surprise de notre part à un vote qui sera très large en faveur de ce gouvernement. De ce projet du gouvernement mais je crois qu'on le doit en partie justement au gouvernement qui avait proposé un projet clair et qui a su convaincre c'est donc nous semble-t-il un aboutissement mérité pour le gouvernement et en particulier pour le ministre. Merci monsieur le président. La parole est à monsieur Jean-Claude Requier.

Madame la présidente, monsieur le ministre. Monsieur le président de la commission des lois, mais si le rapporteur mais j'ai un collègue le 12 août 1789 face à l'Assemblée nationale

si la nécessité d'établir des lois et de les exécuter. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de sécurité mais plutôt de sûreté. Nous parlons de de de sûreté de sécurité plutôt que de sûreté, mais nous chérissons toujours autant de nos libertés et celle-ci ne peut s'exprimer pleinement. Que les, une société qui voit ses règles communes. Nous avons donc aucune pudeur à dire combien le travail de la police et la gendarmerie nationale est précieux. C'est dans cet esprit Que s'est forgé mon opinion sur ce projet de loi de programmation et pour l'essentiel il semble convaincu. Et moyens budgétaires augmentent les perspectives indiqué dans le rapport sont bonnes. Le Sénat a su corriger quelques aspects du texte pour qu'ils sont mieux équilibrés. J'y reviendrai notamment en panne de l'amende forfaitaire délictuelle. Nous avons aussi ajouté certains dispositifs particuliers qui sont les bienvenus. Je pense par exemple par celui de l'article 14 bis. Qui supprime une nécessité de réitération ou de formalisation des menaces de mort pour encourir une sanction pénale ou encore l'article 10 bis qui permettra de reconnaître la qualité d'agent de police judiciaire aux élèves officiers de la reine. Bref, de manière générale, vous vous perdez assure toujours celui les apports de ce projet de loi ce. Cela étant, il a aussi fait des problèmes de réserve. Qui n'ont hélas pas toutes été pleinement dissipé à l'issue de ce travail législatif. Pour point difficile l'amende forfaitaire délictuelle. Les dispositions du projet de loi initial en huit été corrigée par notre hémicycle. Ce fut là justement heureux et nous nous réjouissons de le retrouver dans le texte de la CMP. La des infractions susceptibles de faire l'objet d'une amende forfaitaire est strictement encadrée et mieux encore, il a été pris soin pendant. Renforcer le droit des victimes à préservant la possibilité de se porter partie civile 2ème réserve la suppression de la condition de s'y a noté appliquée aux policiers et gendarmes pour se présenter à l'examen d'OPJ. Nous payons toujours être convaincu, autre groupe croit ou bien jet expérience surtout dans ces métiers où la gravité des décisions et des actes, et parfois vertigineuse. Avait une 3ème. Difficulté, la création d'ailleurs système d'enquête. Sur le principe, nous y sommes ne sont pas hostiles. Cela peut être une bonne chose, mais tout dépendra des modalités de mise en place. Je vois pas quelques-unes des interrogations. Qu'. Mes collègues. Carrère et Nathalie Delattre a au cours de ces de nos des bras. J'ai une. Sur leur formation et leur encadrement. J'ai une. Sur la rue, Libération ou encore des interrogations sur leur répartition. Donc que tout soit fait pour que ce nouveau corps de métier soit effectivement en mesure d'apporter le soutien attendu à la police judiciaire selon ma mère avais à dire un mot de la réforme en cours de notre police. Beaucoup de mes collègues ont relayé les inquiétudes qui entourent ce projet. Certes il y a dans territoire je dirai seulement que la critique n'est pas unanime au cours des certaines auditions.-- J'ai pu des voix en faveur des changements annoncés. Toujours est-il que cette réforme tend à diviser pourrait conduire les ruptures de ce point de vue c'est regrettable Sénat a bien fait de rappeler la nécessaire prise en compte des spécificités de la police judiciaire dans le cadre de la réforme de la relation de la police nationale. Il faut que le gouvernement trouve le moyen de rassurer les agents préoccupé par ces bouleversements à venir ne serait-ce que pour ménager ces hommes et ces femmes qui oeuvrent quotidiennement pour la sécurité de nos concitoyens et le bien public d'automation ces remarques note pas à ce projet de loi, ses qualités que je rappelé mon propos introductif notre groupe, il sera donc très favorable. Merci monsieur le président. Et enfin, la parole est à madame la présidente, Éliane Assassi.-- Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'élaboration du texte donc issu des travaux de la CMP ne nous invite pas à modifier notre position à 7 Lopmi. C'est dommage. Qu'il a bien des égards est un marqueur selon nous des choix politiques qui privilégie le répressif en ignorant la prévention, la dissuasion. En prenant effectivement le tout répressif par la système systématisation de la simplification de la procédure. Je crois que nous ne faisons pas honneur aux professions de la sécurité auquel je suis effectivement très attaché et pour plusieurs raisons, que je n'évoquerai pas ici à cette tribune. Il est intéressant de constater que, selon le ministre de. Le ministère de l'Intérieur. Un policier hyper équipé et non et non un policier de proximité seraient fédérateur et ouvrirait des vocations. Je ne partage pas cet idéal de sur équipement et de répression. Cette conception froide d'missions de nos policiers, nos gendarmes mais également des victimes et des mises en cause n'est pas acceptable sur le plan procédural comme j'ai eu l'occasion de le souligner, nous dénonçons l'extension des autorisations générales de réquisition, la simplification de la procédure pénale induit un affaiblissement des droits de la défense. Une telle autorisation dessert les droits fondamentaux du mis en cause l'imprécision n'est pas au service de la présomption d'innocence ni du droit au respect de la vie privée. La régularité de la procédure pénale risque ainsi d'être remise en cause par de telles réquisitions générale. De plus, la généralisation de l'amende forfaitaire délictuelle à 29 délit privera les justiciables des garanties fondamentales coffre la procédure pénale par un tel procédé la Lopmi déléguera aux agents de police une fonction qui relèvent en principe de l'autorité judiciaire, comme l'a souligné la Cncdh mais également le Conseil d'État dans son avis du 10 mars dernier. Si la commission mixte paritaire agi en toute sagesse, sagesse en limitant la liste des infractions pouvant faire l'objet d'amendes forfaitaires délictuelles, nous aurions je dois dire préféré qu'il ne soit tout simplement pas plus possible d'y recourir. Par ailleurs, l'abaissement des exigences dans le recrutement des OPJ conduira inévitablement à des manquements procéduraux et finalement à des irrégularités qui feront tomber des procédures cette mesure desservira la sécurité que vous promouvez, nous le répétons la responsabilité nécessite l'expérience de même mettre en place la fonction d'assistant de police et de gendarmerie n'est pas un gage d'efficacité. La procédure pénale même dans son aspect le plus infime nécessite vigilance et rigueur. À l'issue de son passage au Sénat et à l'Assemblée nationale, la Lopmi continue de nous présenter une conception je dirais en mode dégradé du fonctionnement de la police. Je souhaite d'ailleurs Monsieur le Ministre vous alerter une nouvelle fois à l'orée de probables mouvements sociaux d'ampleur en réponse au projet de recul de l'âge du départ à la retraite sur la nécessité. J'ai dit de probables. Sur la nécessité de la mise en place d'une nouvelle doctrine de maintien de l'ordre fondé sur l'apaisement et non sur la tension, enfin en ce qui concerne la police judiciaire la Lopmi demeure au l'antichambre de la réforme à venir portant sa départementalisation. Départementalisation synonyme d'intrusion du pouvoir exécutif dans les procédures pénales une nouvelle rédaction de l'alinéa 150 du rapport annexé ne suffira pas à éteindre la colère vive qui s'exprime au sein de la magistrature des barreaux et des enquêteurs de la police judiciaire. Les garanties d'indépendance offerte sont trop faibles. pas à la hauteur des enjeux humains et procéduraux de notre ère, comme en témoigne la décision de la CMP de supprimer l'article 6 bis prévoyant des référents formés sur la lutte contre les discriminations au sein des commissariats et des gendarmeries la CMP brandit le fait que le rapport annexé reprend

être moderne ne se résume pas à se doter d'équipements numériques, être moderne c'est tendre l'oreille agir de façon inventive et demeurer au service de l'intérêt général, par la proximité, la Lopmi n'est pas innovante malgré ses apparences très robotique nous trop donc contre cette cette Merci madame la présidente. Conformément à l'article 42 alinéa 12 du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur le texte élaboré par la CMP. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

ouvert. Ça ne demande à voter. Le scrutin est clos. clos. Voici. Le résultat du scrutin. Nombre de votants 343 exprimés, 343 pour, 316 contre. Contre 27, le Sénat a adopté. Mes chers collègues, je vais lever la séance prochaine séance jeudi 15 décembre à 11h. Pour l'examen du projet de loi de finances pour 2023, en nouvelle lecture. La séance est levée.

Merci